Bonjour mes chers collègues, Monsieur le Ministre, la séance. Est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué, y a-t-il des observations. Je n'en vois pas. Le procès-verbal est donc adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. La parole est à monsieur Jean Bachy, président de la commission mixte paritaire, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, C'est avec une sincère et très vive émotion que je m'adresse à vous ce matin pour marquer l'aboutissement du parcours législatif de ce texte qui a fait l'honneur à l'initiative parlementaire et plus particulièrement aux travaux de notre assemblée. Cette proposition de loi que nous nous apprêtons à adopter définitivement à la suite d'une commission mixte paritaire conclusive est en effet le fruit d'un travail engagé par notre assemblée depuis maintenant un an et demi. Je me réjouis que ce texte est ainsi pu donner une traduction législative aux travaux de la mission de contrôle du Sénat sur l'intensification et l'extension du risque incendie engagé dès le printemps 2022, dont le rapport avait été présenté en août dernier par mes collègues Anne-Catherine Loisier, Pascale Martin, Olivier Reitman et moi même tout au long de nos travaux, nous nous sommes efforcés de tirer des enseignements bien sûr des incendies de l'été 2022 mais aussi de celui de Gonfaron dans le Var en 2021, dont l'intensité nous a malheureusement rappelé l'urgence à agir pour prévenir l'embrasement de nos forêts et plus largement de nos campagnes. Cette proposition de loi a été largement irrigué par les retours de terrain de l'ensemble des acteurs de la défense des forêts contre les incendies, que nous avons amplement entendu. Il s'agit là d'une principale force ne ne ce texte les mesures qu'ils contiennent sont opérationnels et pragmatique et viendront renforcer notre arsenal de prévention et de lutte contre les feux dès cet été. Je ne reviendrai évidemment pas surtout les apports du Sénat sur ce texte, auquel l'ensemble des groupes politiques ont apporté leur contribution mais je retiendrai notamment la création d'une stratégie interministérielle et territoriale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies, l'interdiction de fumer dans les bois et forêts dans un contexte où, rappelons-le, 90% des départs de feux sont d'origine humaine. La consécration au niveau législatif de la possibilité pour les sapeurs-pompiers de réaliser des coupes tactique pour limiter la propagation des feux ou encore l'exonération de l'ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour les véhicules des services d'incendie et de secours qui apportera un coup de pouce financier non négligeable nos au Centre d'incendie et de secours dans un contexte où leurs Budgets sont particulièrement contraignants. Malgré ce satisfecit qui représente une avancée indéniable. Je regrette le caractère inachevé du texte issu de la CMP et au regard d'un certain nombre de propositions que nous avions formulées et qui nous apparaissait comme essentiel. Je laisse pour exprimer cela la parole à notre rapporteur Pascal Martin. Merci monsieur le prix. Dans je laisse donc la parole à monsieur Pascal Martin notre rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire. Chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je prends donc la suite du président Bassy pour exprimer un vif regret le texte que nous vous présentons aujourd'hui n'est pas allé au bout de sa logique sur son volet financier. Il faut dire que nos collègues de l'Assemblée nationale, sous la pression comptable de Bercy ont fait preuve de peu de considération en la matière et plus particulièrement sur 2 mesures phares dans notre proposition de loi, nous avions plaidé pour étendre aux employeurs publics. Le bénéfice de l'article 34 qui prévoyait une réduction de cotisations patronales accordées aux employeurs en contrepartie de la disponibilité de leurs salariés sapeur-pompier volontaire. Nous n'avons pu obtenir gain de cause sur ce point alors que l'inclusion des collectivités locales dans ce dispositif était parfaitement justifiée. Cela est d'autant plus vrai pour les communes rurales pour lesquelles la mise à disposition de leurs employés représente une charge financière non négligeable. Il ne suffira pas de solliciter les employeurs privés pour remédier à la crise du volontariat des sapeurs-pompiers. Les collectivités locales et notamment les petites communes fournissent également un vivier de sapeurs-pompiers volontaires, dont nous nous privons en les excluant du dispositif. Je rappelle qu'il manque à ce jour 50.000 sapeurs-pompiers volontaires sur l'ensemble du territoire métropolitain. J'en viens maintenant à l'article 10 de la proposition de loi qui visait à créer un crédit d'impôt pour les dépenses de travaux réalisés en application des obligations légales de débroussaillement autrement appelé au. Et qui, face à l'opposition de l'Assemblée nationale a dû être retiré du texte final. La création de ce crédit d'impôt aurait pourtant pu provoquer un électrochoc pour inciter les propriétaires forestiers à procéder aux travaux de débroussaillement nécessaires à la protection de leurs habitations dans un contexte où seulement 30% des OL des sont réalisés à ce jour. Face à ce constat implacable, la création d'un tel mécanisme d'incitation à la réutilisation des eaux LD. Aurait été bienvenu, a fortiori pour les propriétaires forestiers les plus modestes. Sur cet article. Mon collègue rapporteur Olivier Reitmans avait pourtant fait preuve d'ouverture en proposant plusieurs solutions de compromis en amont de la commission mixte paritaire finalement restés lettre morte. Il est regrettable que des considérations budgétaires de court terme et pris le pas sur l'objectif de préservation de nos forêts, alors même que les études sur la valeur du sauvé. Je me permets d'insister, montre qu'un euro investi dans la prévention et la lutte contre les feux de forêt en rapporte 20 à 25 fois plus. Je n'ai toutefois aucun doute sur le fait que le projet de loi de finances et le projet de loi de finances, membre de la sécurité sociale 2024. Seront l'occasion pour le Sénat de promouvoir ces mesures et je l'espère, Monsieur le Ministre, que le gouvernement saura faire preuve. De plus, de compréhension dans l'intérêt de nos forêts et nos sapeurs-pompiers, mes chers collègues, le Sénat peut être fier du travail accompli. Les avancées obtenues par cette proposition de loi était attendu, tant par les acteurs de terrain que par l'ensemble de nos compatriotes encore marqué par l'intensité des feux de l'été 2022. Je suis convaincu que les avancées que nous avons obtenu ensemble porteront leurs fruits dès cet été, je vous remercie. Merci monsieur le rapporteur. La parole est à présent à monsieur Franck Riester, Ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Madame la présidente, monsieur le président de la commission. Monsieur le rapporteur. Mesdames, et messieurs les sénateurs. J'ai pris tout d'abord de bien vouloir excuser les absences de Marc Fesneau et Dominique Faure qui sont retenus par d'autres obligations. Permettez-moi, à l'occasion de l'examen de ce texte de rendre un hommage sincère à l'engagement des structures et personnes mobilisées dans la prévention et la lutte contre les incendies de forêt qui vont être remobilisée cet été voir le sont déjà sur certains territoires. Je pense notamment aux Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes et à la Corse. veux remercier une nouvelle fois au nom du gouvernement, tous les acteurs, sapeurs-pompiers, personnels de la sécurité civile. Sapeurs-sauveteurs forestiers sapeurs forestiers qui s'engage pour la sauvegarde de nos forêts et pour l'excellent travail qu'ils effectuent au quotidien. Je tiens également à saluer le travail qui a été effectué par l'ensemble des parlementaires pour aboutir à un accord en commission mixte paritaire. Si les incendies ont toujours existé leur intensification nécessite une action conjointe du Parlement et du gouvernement et je me réjouis que sur ces sujets. Un travail de coconstruction puisse se faire dans de bonnes conditions. En effet, le climat change les incendies hors norme de l'été 2022 générée par un concours de sécheresse et de températures particulièrement élevées ont apporté la preuve éclatante et douloureuse des effets à attendre du changement climatique en matière de feux de forêt. Il laisse entrevoir une intensification du risque dans les régions historiquement concernés du Sud-Est du Sud-Ouest et de la Corse mais aussi. Et surtout une extension du risque dans des régions jusqu'ici préservé. Je pense notamment aux régions de l'Ouest de l'Est et du centre de la France territoires dans lesquels nous n'avions pas vu d'incendies de cette ampleur auparavant. Notre politique de prévention et de lutte contre ces incendies doit donc être renforcée et actualisée au regard d'un risque amplifié étendu sur davantage de territoire. Nos concitoyens attendent des réponses rapides et concrètes à leurs inquiétudes lorsqu'ils voient les incendies parcourir de si grande superficie de forêt sur l'ensemble du territoire national. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sur ce texte et de l'inscrire sur son ordre du jour à l'Assemblée nationale afin qu'il chemine rapidement jusqu'au terme de la navette parlementaire. Le prion de la République a annoncé en octobre dernier, plusieurs mesures visant à renforcer notre politique nationale de défense des forêts contre l'incendie. Tout d'abord la prévention demeure essentielle bien sûr notre stratégie et d'éviter le départ de feu et d'être en mesure d'attaquer les feux naissants, pour éviter leur propagation. Des moyens supplémentaires ont ainsi été. Cette année par mon collègue Marc Fesneau à l'Office national des forêts pour lui permettent de renforcer ses missions de surveillance et de première intervention et de les étendre dans des territoires nouvellement concernées par ce risque. Des moyens supplémentaires ont également été apportées à l'association régionale de défense des forêts contre les incendies des Landes de Gascogne massif riche d'une organisation impliquant les propriétaires forestiers ce renfort de moyens se poursuivra en 2024. Mais il va falloir davantage agir sur l'origine des feux. Lorsqu'on sait que 90% des départs de feux de forêt sont liés à une activité humaine. Notre priorité est d'intervenir sur les interfaces entre forêts et habitations. Soyons clairs, les obligations légales de débroussaillement fixés dans le code forestier doivent être mieux mises en oeuvre alors qu'on estime qu'elles le sont seulement à hauteur de 30% à ce jour. Pourtant, leur efficacité n'est plus à démontrer. Nos moyens de lutte doivent impérativement être renforcé pour limiter la propagation des feux ensuite protéger nos concitoyens et sécuriser nos infrastructures lors des débats dans cet hémicycle le sujet de la prévention a été longuement débattue. Et de nombreuses avancées ont été voté en ce sens. Toutefois, malgré tout ce que l'on peut faire le feu arrivera. La lutte doit donc également être mieux organisé, le président de la République ainsi décide de renforcer les moyens terrestres, aériens dédié dès cette année. Je tiens d'ailleurs à saluer la reconnaissance dans ce texte du caractère dangereux du métier des missions exercées par les personnels navigants de la sécurité civile comme la loi le fait déjà pour les sapeurs-pompiers professionnels depuis 2004. Cette reconnaissance symbolique était nécessaire, alors que l'ampleur de leur tâche ne cesse de grandir. Enfin, nous sommes loin de tout savoir sur l'évolution de ce risque. Nous avons ainsi missionné nos inspections générales pour actualiser la cartographie du risque incendie et nous permet de définir nos organisations cibles pour y faire face dans les années à venir. Les conclusions de cette mission seront connus cet été et nous permettront de nous préparer pour l'année prochaine et bien sûr les années suivantes. Ce texte est donc plus que bienvenue. Il propose en 1er lieu l'inscription dans la loi d'une stratégie nationale et interministériel de défense des forêts contre l'incendie qui permettra de mobiliser pleinement et largement l'ensemble des acteurs concernés, public et privés. La task force interministérielle déjà mises en place par le gouvernement sera missionné pour l'élaborer et organiser les concertations nécessaires. Le texte propose également de faire évoluer la liste des territoires réputé particulièrement exposés aux risques d'incendie. Ce qui permettra d'être plus réactifs face aux évolutions du changement climatique. Cette liste doit aussi nous permettent d'assurer un déploiement efficace de nos moyens de prévention et de lutte vers les territoires reconnus comme les plus exposés en outre le texte suggère d'améliorer l'articulation des mesures de défense des forêts contre l'incendie avec les autres politiques publiques, notamment celle des sites classés et de protection de l'environnement ce qui renforcera la cohérence et de lisibilité de nos actions pour nos concitoyens. Concernant la politique de l'urbanisme justement je salue les propositions pour améliorer l'information du grand public, des élus locaux et des futurs acheteurs sur la sensibilité aux dangers prévisible des feux de forêt et de végétation. Je pense aussi au monde agricole qui a des solutions à apporter que nous devons reconnaître et accompagné notamment les coupures agricoles lorsqu'elles sont judicieusement positionnée. Par ailleurs, comme je le disais précédemment, les obligations légales de débroussaillement sont essentiels à mettre en oeuvre et le texte prévoit des clarifications et simplifications utiles et attendus pour améliorer significativement leur mise en oeuvre. Je salue aussi la reprise dans ce texte de 2 évolutions issues des Assises de la forêt et du bois, à savoir l'abaissement à 20 hectares de l'obligation de disposer d'un plan Simple de gestion et la systématisation de la télé-déclaration. La mise en place d'un document de gestion durable est en effet la première étape permettant à un propriétaire de connaître et de maîtriser les risques pour sa forêt. Par ailleurs, l'inscription dans la loi d'une journée nationale de la résilience permettra de mieux nous a culture et collectivement aux risques naturels, notamment ceux liés aux effets du changement climatique. Le texte comprend enfin des dispositions importantes pour les sapeurs-pompiers volontaires et les services départementaux d'incendie et de secours. Il prévoit notamment à titre expérimental une exonération d'une partie des charges patronales pour les entreprises qui libéreront des sapeurs-pompiers volontaires pour aller en opération. C'est une avancée importante pour favoriser la disponibilité, la mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires. En conclusion, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs les sénateurs. Cette proposition de loi est un signal fort envoyé aux propriétaires forestiers aux riverains des forêts aux associations de protection de l'environnement, aux élus locaux et à tous ceux qui s'engagent au quotidien dans la prévention et la lutte contre les incendies de forêt. Ils leur montrent que nous sommes capables d'avancer ensemble pour mieux nous adapter au changement climatique. Je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, je rappelle qu'en application de l'article 42 alinéa 12 du règlement, le Sénat examine après l'Assemblée nationale, le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le gouvernement en conséquence le vote sur l'amendement et sur l'article est réservé. Nous passons à la présentation de l'amendement du gouvernement avant d'en venir aux explications de vote par groupe. Amendement numéro un monsieur et et unique, monsieur le ministre, de coordination, madame la présidente. Quel est l'avis de la commission. Monsieur le rapporteur. Avis favorable. Parfait vote donc réservés. Nous passons aux explications de vote, des groupes à raison d'un orateur par groupe. La parole est à présent à madame la présidente, Éliane Assassi, du groupe communiste et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre planète brûle jamais citation n'aura été si vrai c'est pourquoi. nous saluons les travaux de Madame Loisier ainsi que des rapporteur de cette proposition de loi après de près de 72 articles. Les méga feux de l'an dernier ont emporté près de 70.000 hectares de forêt, ils appelaient à une action du législateur Cévennes Gironde du Rhône mais aussi Bretagne aujourd'hui aucun de nos massifs forestiers n'est à l'abri. C'est une alerte, une traduction concrète du changement climatique. bien que la saison des feux n'est pas encore commencé, 1000 hectares ont déjà brûlé en avril à Cerbère dans les Pyrénées-Orientales. C'est pourquoi. Nous accueillons favorablement ce texte qui vise à renforcer la capacité de l'État et de ses services de la sécurité civile et de la population à prévenir et à lutter contre le risque incendie en posant les bases d'une stratégie nationale interministérielle en abaissant le seuil d'élaboration des plans simples de gestion dans les forêts privées ou encore en imposant l'élaboration d'une carte d'aléa pour cartographier le risque d'incendie. Nous partageons également le renforcement de la sensibilisation, sensibilisation des citoyens, élus et professionnels concernés de même. Nous saluons le renforcement des sanctions en cas de non respect des obligations de débroussaillement en effet la question des zones d'interface habitat forêt est essentiel car dans ces espaces le risque de départs de feu est élevé et La difficile protection par les pompiers et coûteuses. à peine 30% d'entre elles sont réalisées. Pourtant si les départs de feu sont souvent le fait de comportements humains. L'assèchement de la végétation sous le soleil brûlant facilite les départs, puis le développement de ces feux. En ce sens, le respect des eaux Elder est un élément majeur de politique de prévention et à cet égard, il serait opportun que les communes bénéficier de dispositifs d'accompagnement, y compris financiers pour faire face à leurs obligations. Toutefois malgré des progrès indéniables, ce texte ne propose pas de changement de modèle dans notre approche de la forêt et sa multifonctionnalité via un plan plus général d'adaptation de la forêt aux changements climatiques afin de permettre à la forêt française de jouer pleinement son rôle dans l'atténuation du réchauffement et de ses conséquences. Il nous faut investir dans une politique forestière forestière préventive qui permettra la résilience de nos forêts, à commencer par la diversification des essences les forestiers doivent renouveler les peuplements dépérissant et adopter et adapter les forêts françaises en tenant compte des risques futurs. De plus. Les moyens restent en deçà des besoins, que ce soit pour l'ONF qui a perdu plus du tiers de ses effectifs en 20 ans alors qu'il gère près de 25% de la forêt métropolitaine. De 16.000 salariés que comptait l'Office en 1986. Il ne reste plus que 8400 aujourd'hui, auquel l'État continue pourtant de confier à un nombre équivalent de mission et exige une grande rentabilité pour le STIF. Le Centre national de la propriété forestière ou encore météo France même problématique tous manque de moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Toujours en matière de moyens les sapeurs-pompiers souligne entre autres exemples, l'insuffisance du parc de camions citernes feux de forêt ils chiffrent les besoins à 10.000 camions. Ils en ont 3700 actuellement avec un coût unitaire de 300.000 euros, un tel investissement est impossible pour les SDIS. De même, comment oublier que côté renouvellement de la flotte aérienne le 1er Canadair n'arrivera pas avant 2028, alors même qu'en 2010 déjà, un rapport de la mission interministérielle sur le changement climatique et l'extension des zones sensibles au feu au feu de forêt préconisé un moyen à un renforcement des moyens aériens, la dimension de la flotte n'a pas augmenté depuis les années 80 alors que le risque hier circonscrit au pourtour méditerranéen s'est étendue à l'ensemble du territoire et tout cela, tout cela c'est le résultat de politique austéritaire aveugle à la réalité, c'est le résultat de décisions politiques comme celle par exemple que le gouvernement a, en 2020. Quand quand le gouvernement en 2020, à retirer le soutien de l'État aux dépenses d'investissements des SDIS et malheureusement ce texte n'y remédier. Ni remède dira pas. Cela dit, malgré ces réserves, nous voterons le texte de la CMP.

Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, à peine plus d'un an se serait donc écoulé entre le lancement de la mission sénatoriale sur la prévention des feux de forêt et la promulgation, nous l'espérons très prochaine des dispositions de cette loi d'initiative n'a ce la sénatoriale. Adopté à l'unanimité au Sénat et je veux vraiment saluer l'engagement de tous nos collègues de surtout de tous les groupes sur cette PPL face à l'importance des enjeux. Nous nous réjouissons tous ceux que l'objectif d'une loi opérationnelle avant la saison des feux et pu être tenu. La version finale de cette loi dont la logique, je le rappelle, s'inscrit dans une adaptation continue de notre politique de prévention des feux en fonction de la, de l'évolution de l'aléa conserve la majeure partie des propositions initiales de notre rapport sénatorial l'élaboration d'une stratégie interministérielle et territoriale de nouveaux outils de régulation entre la forêt et ces interfaces avec les zones habitées et les infrastructures et notamment le sujet des eaux S'agissant du volet forestier notre rapport d'information préconisé une forêt mieux gérer pour être moins vulnérable aux risques au risque que le feu se développe avant d'être détectés risquent de ne pouvoir accéder au feu faute de desserte aménagé et et entretenu risque de progression rapide de l'incendie, alimenté par une masse combustible au sol. L'accord trouvé en CMP préserve ses dispositions combinant Prog'progrès des pratiques et accompagnement de la filière il dessine ainsi au final une loi équilibrée a même nous le pensons, de répondre à l'extension du risque sont ainsi mis en place des financements publics destinés à l'amont forestiers notamment au reboisement qui seront ma chère collègue assujettis à une et conditions éco-conditionnalité et une conditionnalité DFCI par exemple en termes de diversification de respect des zones pare-feu afin de ne pas répéter les erreurs du passé le seuil à partir duquel il sera obligatoire pour un propriétaire forestier de se doter d'un plan simple de gestion passe de 25 à 20 hectares emportant ainsi 500.000 hectares supplémentaires dans la gestion durable. Parallèlement le risque incendie est intégré de façon plus cohérente dans les documents Cadre de la politique forestière. Nos communes pourront faire valoir dans des conditions encadrées, un nouveau droit de préemption DFCI sur des parcelles boisées non. Se situant au milieu d'un couloir de feu afin de prévenir le risque par une gestion forestière plus plus adapté. Le taux réduit de TVA pour les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière est également prorogé de 2 ans jusqu'en 2025 et enfin dans une même logique et afin de susciter des travaux de gestion en forêt le périmètre du dispositif DEFI-Forêt être étendue aux 24.000 petite propriété boisée et aux 210.000 hectares dotés de ce que l'on appelle des codes de bonnes pratiques sylvicoles plus c'est-à-dire avec programme de coupe et travaux. Au-delà de ces réels progrès acté demeure tout de même et ça été évoqué des points déterminants sur lesquels nous n'avons pas pu aboutir, tout d'abord les députés n'ont pas voulu faire figurer dans la loi de puissants leviers financiers nous privant d'outils opérationnels majeurs pour aider les collectivités et les particuliers à faire face au risque incendie ainsi les collectivités mettant à disposition du se disent leurs salariés ne pourront pas être soutenus financièrement par le biais d'exonérations de charges. De même, les particuliers, et singulièrement les plus modestes qui sont confrontés à des coûts de premières obligations légales de débroussaillage élevé ne pourront pas être aidés par un crédit d'impôt incitatif. Autre point en suspend le financement de la présence humaine supplémentaires préconisés par la loi est nécessaire sur nos massifs forestiers pour l'ONF l'hémorragie a été stoppée lors du dernier exercice budgétaire mais il faudra renforcer les effectifs sur le terrain. Quant aux missions supplémentaires que nous confions au Centre national de la propriété forestière que vous avez salué Monsieur le Ministre, elles appellent la création d'une trentaine de postes temps pour constituer le réseau des référents DFCI prévu par la loi que pour prendre en charge le flux important des nouveaux documents de gestion durable qui seront mises en place avec cette loi, que le groupe centriste soutiendra. Nous sommes donc à l'aube de nouvelles adaptations de notre organisation DFCI les règles et les principes fixés se mettront progressivement en place en place sur les territoires et contribueront à construire cette nécessaire culture du feu partout dans l'Hexagone. Notre rôle de législateurs sera de veiller avec soin à la bonne application de ce texte en revenant dès cet Automne et dès le PLF sur les manquements et les ajustements financiers nécessaires à son efficacité. Je vous remercie. Merci cher collègue. La parole est à présent au sénateur André gris Guillaume pardon du groupe RDSE. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Merci madame la présidente. Monsieur le Ministre. Monsieur le président de la Commission, mon cher Jean. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Renforcer la prévention et la lutte contre les incendies de forêt est devenue aujourd'hui une impérieuse nécessité. En 2022, l'Europe a dû faire face à une niveau record de surfaces brûlées par des feux de forêt. Plus de 785.000 hectares, soit plus du double de la moyenne enregistrée un taux 6 2021. Nous ne pouvons pas dans le cas de cette PPL ne pas évoquer aussi la les gigantesques et dramatique, un syndicat d'Indiens qui viennent impacter notre atmosphère et qui demain probablement perturberont encore plus le climat planétaire. J'en profite pour saluer l'intervention de nos sapeurs-pompiers qui sont allés prêter main forte à leurs collègues et nos amis canadiens. Mon département le Var n'est hélas pas épargnée par les feux de forêt et ce depuis longtemps. Un territoire largement couvert par la forêt par ses collines mais aussi une région confrontée à une sévère sécheresse. Les prévisions météo de cet été 83 annonce une saison encore plus chaude que d'habitude. Et si le mistral fait son apparition. Nous craignons de devoir affronter une période encore plus critique. En Côte d'ailleurs en ce début de ces zones déjà plusieurs départs de feu comme à Grimaud et à Carqueiranne que la politique de prévention et de vigilance de nos comités communaux de feux de forêt couplée avec la réactivité des sapeurs pompiers ont pu maîtriser. Il fallait donc s'armer de tous les moyens nécessaires pour faire face à ces crises récurrentes et en voie d'intensification des moyens humains, matériels et juridiques. Certes le Sénat n'a pas attendu pour se mobiliser puisque nous nous étions déjà engagés dans des travaux relatifs à la lutte contre les incendies au moyen d'une mission de contrôle. Je tiens donc à saluer. Nos collègues. Anne-Catherine Loisier. Bassi. Pascale Martin et Olivier. Pour leurs investissements à la hauteur de ces enjeux. Car il devenait impératif d'élaborer une stratégie nationale interministérielle de lutte contre les incendies. Tout comme nous devions poursuivre nos efforts afin de mieux réguler les interfaces. Zone urbaines de dynamiser respectueusement de la biodiversité, la gestion forestière tout hein sensibilisant davantage les populations au risque incendie. Ce texte doit marquer une meilleure prise de conscience de notre nation face aux catastrophes qui s'intensifie, année après année. Je me réjouis que les 2 assemblées donc su trouver un accord en CMP sur un sujet aussi fondamental que notre sécurité pour la sauvegarde des biens pour la préservation de l'Aviron ne manquent confrontés au défi climatique. Cette proposition de loi, l'illustrent bien. Nos institutions et tout particulièrement le Sénat se sont donc mobilisées pour créer de nouveaux outils et renforcer ce qui existait déjà. Le résultat est imposant avec initialement 38 articles nous en arrivons aujourd'hui à plus de 70 révélateur que ce texte n'est pas juste un affichage politique mais bien un travail de fond. Détaillée et approfondie. J'en profite aussi pour saluer l'importante contribution dans ce contexte De notre collègue Nathalie Delattre sénatrice de Gironde également concernés par ces sinistres et dont les travaux resteront. Imprégnée dans cette loi bientôt adopter je pense en particulier au renforcement du rôle des associations syndicales autorisées de DFCI dans l'ensemble du texte notamment en vue d'élaborer une stratégie nationale interministériel de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies. il demeurera aura également son amendement adopté par notre assemblée concernant l'ajout de coupe tactique et parmi les méthodes de lutte contre samedi auquel peut recourir le commandant des opérations de secours. Regrettons cependant et ça vient d'être dit que la suppression du crédit d'impôt pour la défense pour la dépense des travaux réalisés en application des obligations légales de débroussaillement notamment sur les terrains voisins des zones naturelles, ce qui aurait été un outil efficace. Rappelons qu'en vue d'établir une véritable stratégie nationale cohérente, la nécessité de disposer d'une 4ème, unité d'intervention et d'instruction de sécurité civile qui serait situé dans le sud-ouest du pays, du pays, une unité identiques à celles de Brignoles de Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loir et de Corté comme l'a annoncé le président de la République le 28 octobre 2022. Après les terribles feux de forêt de Gironde de la de toutes ces considérations. Cette proposition de loi est une véritable avancée dans le domaine. Gageons qu'elle sera à la hauteur des attentes. Vous l'aurez compris, mes chers collègues. Notre groupe RDSE votera unanimement en faveur de cette proposition de loi, je vous remercie. Je vous remercie, cher collègue. Merci de vos mots aussi. La parole est à présent à monsieur Laurent Burgo a du groupe les républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale. Monsieur le rapporteur. Mes chers collègues. Le 4 avril dernier nous adoptions ici-même à l'unanimité cette proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie. Il s'agit là d'un texte issu d'un travail important. Sénatoriales, fruit de recommandation d'une mission de contrôle. Élu d'un département particulièrement concerné. Permettez-moi de saluer le travail là. L'investissement de nos collègues, monsieur le président jamais assis et des rapporteurs Anne Katerine Loisier Pascale Martin et Olivier Rickman. Mieux vaut prévenir que guérir. Voilà un adage de bon sens qui s'applique également en matière de risque incendie. Les feux hors norme de l'été 2022 et la sécheresse de ces derniers mois n'ont fait que confirmer l'urgence à agir pour prévenir l'embrasement dans nos forêts. À l'issue de la commission mixte paritaire qui nous a réunis le 19 juin dernier nous avons su préserver des avancées notables sur des mesures stratégiques et surtout opérationnel. Nous pouvons ainsi nous féliciter de la mise en place de nouveaux outils de régulation entre les espaces forestiers et les zones habitées et ce par la clarification des obligations légales de débroussaillement dites Walder ou encore avec les surfaces agricoles. Notons également plusieurs aides fiscales l'exonération de TICPE c'est-à-dire de la taxe sur le carburant pour les véhicules des services d'incendie et de secours, ce qui pour les coïncide. Qui nous regardent devait être une aberration. En fait, notons l'extension du dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement. À 24.000 petits propriétaires. Nous pouvons également nous réjouir de la mise en place contre les incendies d'une stratégie interministérielle et territoriale de défense des forêts, mais aussi des surfaces non boisées soulignant encore la mise en place d'un cadre réglementaire adaptable ainsi qu'une intégration plus cohérente du risque incendie dans la gestion de nos forêts. Néanmoins, et comme souvent lors d'âpres négociations les avancées acquises sont aussi teintée de regrets, mais sans remords. Monsieur le Ministre, en effet. Ne pourrait être déçus de l'absence. Le texte final de de mesures. 2 mesures auxquelles le Sénat était attaché et pour lesquels nous avons bataillé jusqu'au bout et se disons-le. Malgré une attitude peu constructive de nos collègues de l'Assemblée nationale, alors même que nous leur album proposé plusieurs comme promis. Un défenseur des collectivités territoriales. Nous regrettons l'exclusion de ces dernières du dispositif de réduction des cotisations patronales accordées en contrepartie de la mise à disposition d'employés sapeur-pompier volontaire. N'hein des collectivités et notamment les communautés les communes rurales pour lesquelles était la mise à disposition constitue une charge non négligeable. La sécurité civile se privé d'un vivier considérable de sapeurs-pompiers volontaires au nom de considérations budgétaires coût termistes. Je rappelle que les études sur la valeur du sauver moindres que un euros investi dans la prévention et la lutte contre les feux de forêt en rapporte 20 à 25 fois plus et il faudrait peut-être que Bercy comprennent cela. Enfin pour le gardera que je suis. Il a été difficile de prendre acte du retrait dans le texte du crédit d'impôt pour les dépenses réalisées en application des obligations de débroussaillement ces fameuses OL La création de ce crédit d'impôt adopté à l'unanimité par le Sénat aurait provoqué un électrochoc pour inciter les propriétaires à les réaliser. Je tiens à le rappeler ici, d'autres l'ont fait au préalable. Seulement 30% d'entre elles sont aujourd'hui respectées, alors même que leur efficacité n'est plus à démontrer. Bien sûr il peut parfois s'agir d'irresponsabilité mais croise un des témoignages reçus lors de mes déplacements dans le Gard. Il s'agit bien plus souvent soit d'une ignorance de la réglementation en elle-même, soit bien plus couramment d'un manque de moyens. D'ailleurs, qu'il ne vaudrait pas mieux protéger son domicile contre les incendies. Alors oui, ce crédit d'impôt et constituer un vrai coup de pouce à l'égard des foyers les plus modestes et pour lesquelles ces travaux représentent exclusivement qu'un coût bien trop élevé. De nature optimiste. Il faut bien, j'aime à croire que les graines que nous avons planté au cours de cette navette parlementaire puisse prochainement porter leurs fruits, notamment lors des débats de l'Automne prochain autour du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. En tout cas nous serons au rendez-vous en conclusion. Mes chers collègues. Malgré ses regrets. Oui avec mon groupe nous voterons ce texte car, comme le formuler, l'abbé Pierre. On ne peut pas, sous prétexte qu'il est impossible tout faire un jour. Ne rien faire du tout. Je vous remercie. La parole est à présent à Madame Vanina Paoli-Gagin du groupe les indépendants et vous avez 5 minutes. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en avril dernier en première lecture de ce texte j'introduisait mon propos en alertant sur le fait que l'été passé serait malheureusement notre avenir. Il est même notre avenir immédiat. Notre sécheresse estivale s'est transformé en sécheresse hivernale les violents feux de forêt cet été en tristement cédé la place aux feux de cet hiver. Nous ne cessons de le répéter, plus aucun territoire n'est épargné. L'adaptation n'est plus une option, c'est une urgence. Plus aucun citoyen ne peut. Se sentir autrement que concernés par ce défi majeur. La prévention est l'une des pièces maîtresses de la lutte contre les incendies. Enfin, nous sommes tous conscients qu'une réaction appropriée avec des outils renouvelés. Agile et efficace et nécessaire. Le triptyque adaptation prévention réaction à guider nos travaux et je m'en réjouis. Je note que le texte a presque doublé de volume entre son passage au Sénat et son étude à l'Assemblée nationale. Si je pense que nous avions besoin de réformer en profondeur notre système. Je m'interroge, mes chers collègues, tout de même quant à l'inflation normative. De manière générale et en particulier sur ce texte. Si nous voulons gagner en efficacité déployé les 3 grands axes que je viens de citer, nous devons avoir des règles claires. Facile à mettre en place. Nous oublions souvent que nos lois manque de praticité c'est pourtant primordial pour ceux qui les appliquent au jour le jour. Je pense à nos élus, ainsi qu'à nos combattants du feu et notre sécurité civile dans sa globalité. Quand il s'agit du risque incendie chaque minute compte des outils trop complexe ne peuvent constituer un frein. Je salue les travaux préparatoires sous la houlette d'Anne-Catherine qui ont, qui nous ont menés au Sénat à la discussion de cette proposition de loi et à la construction législative que nous avons aménagé. Je me félicite que nous soyons arrivés rapidement à un accord sur ce texte il est équilibré. Le voleur réglementaire. Monsieur le ministre devra intervenir très rapidement. Les annonces faites depuis le 28 octobre dernier me sans aller dans le bon sens. Les préconisations du rapport sur la modernisation de la sécurité civile et la protection contre les risques majeurs seront sûrement des pistes de réflexion intéressante pour poursuivre notre travail. Déjà le renforcement des moyens financiers et matériels et humains est une bonne nouvelle, le fonds vers les informations délivrées aux élus, aux propriétaires et aux citoyens sont une étape essentielle. Je salue à cet égard comme cela a déjà été fait par mes collègues la météo des forêts introduite par météo France savoir c'est effectivement pouvoir anticiper et notre vigilance via ce type d'outils et renforcée. En première lecture. J'avais évoqué la sensibilisation des citoyens et des propriétaires. À la fois sur les interdictions de fumer aux abords et dans les forêts qui doivent devenir un réflexe, le même que celui de mettre notre ceinture de sécurité lorsque nous montons dans un véhicule. Il en va de même pour les obligations légales de débroussailler. L'un des points centraux de notre proposition de loi. Je me réjouissais en avril dernier de voir pérenniser le défi que nous avions déjà prolongé lors du dernier projet de loi de finances. Le texte de la CMP propose de le prolonger à nouveau jusqu'en 2027. Nous devrons remettent néanmoins ce point sur le métier et resteront vigilants. Nous avons bien observer le rôle décisif des agriculteurs dans la lutte contre les incendies. Je trouve ainsi tout à fait logique de les associer à différentes étapes. Notamment via les champagnes d'agriculture sur les plans de protection et de prévention. De plus, l'inclusion des surfaces agricoles dans la lutte contre les incendies marque la connaissance de la complexité de notre territoire. Cette proposition de loi est tellement riche, mes chers collègues, que je ne pourrais bien évidemment pas évoquer tous ces points, comme celui concernant les mesures visant les salariés sapeur-pompier volontaire que je trouve facilitatrice. Cependant je souhaite clôturer mes propos en vous disant qu'il reste encore beaucoup à faire. Malgré le travail déjà fourni. Je crois particulièrement important sous un angle. De travailler sur le morcellement de nos forêts. Nous le faisons dans l'Aube, notamment sous la houlette du PETN Otar Armand s'pour reprendre la main sur nos forêts et parcelle de forêt, qui sont bien sans maître ou abandonnés. C'est effectivement aujourd'hui une faiblesse dans notre système, faisant une force c'est aux élus locaux et un au législateur de trouver des solutions adaptées. La forêt souffre elle est pourtant l'un de nos meilleurs alliés dans la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité. Les dernières nouvelles sont alarmantes dans le Grand-Est, d'où je suis l'élu dans l'Aube, nos forêts commencera à émettre du CO2. Ce texte est un espoir mais ne nous trompons pas, mes chers collègues, l'action doit se poursuivre. Le groupe les indépendants votera unanimement en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à madame Monique de Marco du groupe des écologistes et vous avez 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre. Madame la rapporteure messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Chaque jour, l'actualité nous rappelle la menace que fait peser une intensification du risque d'incendie sur nos territoires. Alors que la saison des feux commence à peine. Le Canada a déjà perdu plus de 7 millions d'hectares de forêts. Les feux ont pris une telle ampleur que la fumée des incendies chargé en particules fines est arrivé jusqu'en France. Je tiens à apporter tout mon soutien aux soldats du feu canadiens et internationaux qui se battent sans relâche pour stopper ces feu. Cette catastrophe doit résonner dans cet hémicycle comme une alerte ce ce que deviendra bientôt la norme. L'été dernier, plus de 7007, 1000 hectares dont sont partis en fumée. L'été 2022 a été en Gironde très traumatisant. Les climatologues considère que ces canicules ces sécheresses et ces incendies préfigure les étés futurs. Dans son rapport sur les feux de forêt. Le changement climatique. L'OCDE rappelle que l'occupation des sols, la dégradation de l'environnement et les dérèglements climatiques sont en partie responsables de ces catastrophes. Face à l'inaction. Ce même rapport appelle à accélérer la lutte. Contre le changement climatique pour limiter des coûts économiques sociétaux et environnementaux des incendies. Pourtant, alors que nous devons nous préparer à des feux plus nombreux plus étendue et plus violents. Le texte que nous étudions aujourd'hui malheureusement fait l'apologie des petits pains. Certes les moyens supplémentaires déployés en France pour faire face à l'été 2023 dans le bon sens en Gironde le prépositionnement d'avions Air Tractor d'un Dash d'un hélicoptère répond en partie aux besoins immédiats. Les engagements pris par le ministre de l'Intérieur pour envisager la création d'une seconde baisse de Canadair sur la façade ouest sont également positifs. Par contre lors de la commission mixte paritaire. Le gouvernement assumé son manque d'ambition en se limitant des considérations budgétaires. Ce texte n'est plus qu'un petit texte regroupement de petites mesures aux répercussions limitées. Alors qu'il manque 50.000 sapeurs-pompiers volontaires en France. Exclure les collectivités locales au du dispositif de réduction des cotisations patronales est un non-sens sens. Même des mesures évidentes, comme la prise en compte des besoins de la sécurité civile dans la politique de gestion de l'eau ont été supprimés. Pourtant, il s'agit d'une demande nous sapeurs pompiers qui s'inquiètent de la rue de l'avenir en la ressource en eau. Alors que 95% des départs de feux sont d'origine humaine. La sensibilisation de nos concitoyens. Bon réflexe est un enjeu majeur. Prévenir le risque d'incendie passe aussi par la réduction des départs de feu. Malheureusement les mesures proposées dans ce texte sont bien maigre au regard de l'enjeu. Nous avions déjà soulevé cette faiblesse en avril dernier. Mais suite à la CMP de résultats encore plus nette et décevant. Nous regrettons également, comme certains de mes collègues la suppression du crédit d'impôt pour la réalisation des obligations légales débroussaillement adopté à l'unanimité au Sénat. Pour prévenir le risque et sensibiliser la population, nous devons nous satisfaire d'une journée nationale de la résilience à défaut des moyens, nous aurons des paroles. Enfin, l'adaptation de nos forêts au dérèglement climatique est le parent pauvre de cette petite loi. Prévenir le risque c'est également préparer nos forêts aux chaleurs extrêmes aux sécheresses à répétition et aux attaques parasitaires. Augmenter la résilience de nos forêts, c'est réduire le risque d'incendie, c'est soutenir nos sapeurs-pompiers une collectivité, c'est protéger nos concitoyens. Pourtant, les rares avancées que nous avions obtenu au Sénat et à l'Assemblée nationale ont été balayés lors des CM L'absence de mesures en faveur de la biodiversité, nous inquiète. La suppression de la mention biodiversité dans les plans cinq de gestion n'est pas anodine. L'industrialisation de la forêt. Les monocultures et le court-termiste ne font qu'accroître le risque d'incendie. Il suffit de regarder la campagne de replantation en Gironde. Malgré les aléas des chercheurs ont replanter du pin maritime à perte de vue. Les considérations financières ont pris le dessus sur l'objectif de cette loi. Comme l'a précisé Monsieur Pascal Martin, d'autres collègues. Un euro investi dans la lutte contre le feu de forêt génère 20 à 25 euros d'économies en valeur du. Mieux vaut prévenir que guérir. Tout le monde connaît ce proverbe. Hier, lors de la présentation du rapport du Haut Conseil pour le climat. La présidente a jugé que la France a été dépassée par les événements climatiques extrêmes qui l'ont frappé en 2022. Elle appelle le gouvernement à acter l'urgence il a accéléré son action. Elle considère que c'est peut-être la fin des petits pas mais pas encore le pas de courses. Alors oui, mes chers collègues. Le groupe écologiste solidarité et territoires malgré nos et réserve, il y à contrecoeur, nous voterons ce texte. Il s'agit d'une occasion manquée. Pour enfin apporter une réponse à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. Merci la parole est à présent à Madame. Patricia Schillinger du groupe RDPI. Et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous avons tous à l'esprit les images de cet été ou 72.000 hectares de nos forêts sont partis en fumée et avec eux, autant d'hectares de notre Patrimoine naturel. Je tiens à remercier les sapeurs pompiers qui ont lutté jour et nuit contre ces feux de forêt dans mon seul département du Haut-Rhin, ce sont 500 départs de feu recensés en 2022 sénatrice d'une région frontalière. Je tiens à rappeler que l'été dernier, nous avons pu compter sur l'aide de nos partenaires européens avec l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne permettant de mobiliser 4 avions de la flotte Rescue. Le caractère hors norme de l'été 2022 ne doit pas cacher le fait que l'intensification des feux de forêt éteint mon mouvement de fond sur le pourtour méditerranéen français. Les surfaces brûlées pourrait augmenter de 80% d'ici à 2050. Les conséquences du changement climatique se manifestent de manière spectaculaire à l'horizon 2050 50%, des Landes et des forêts métropolitaine seront exposés à un risque d'incendie élevé contre un tiers, il y a un peu plus d'une décennie. La période à risque devraient également être 3 fois plus longue et les feux hivernaux vont se multiplier dès le mois de mai 2022, le Sénat s'est saisi de ce sujet en constituant une mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l'intensification et l'extension du risque d'incendie à l'origine du texte que nous examinons aujourd'hui je veux ici remercier très sincèrement les rapporteurs je tiens à m'associer aux propos de Pascal Martin sur l'article 32 et 34, les travaux de cette mission. Ont mis en lumière la le constat de la future vulnérabilité de notre stratégie de lutte contre le feu de forêt qui elle reste aujourd'hui un modèle de l'Europe qui doit évoluer sans changement notre stratégie de lutte ne suffira pas. Face à l'intensification de l'extension des feux de forêt. La proposition de loi qui en a résulté profond pour partie à cette nouvelle problématique en mettant l'accent sur l'aménagement du territoire, la gestion durable la valorisation de la forêt. La mobilisation de l'ensemble des acteurs au 1er rang desquels les agriculteurs maillon essentiel dans l'élaboration de du modèle de lutte contre les feux de forêt au XXIe siècle demi-depuis 2017 nous avons investi de manière conséquente dans la sécurité civile, avec une autre budgétaire de 40% et l'acquisition de nouveaux avions Dash, force est de constater que la mobilisation de moyens financiers ne suffira pas pour répondre à l'intensification de la presse pression qui s'exerce sur nos massifs forestiers. C'est pourquoi nous avons clarifié le cadre d'intervention des SDIS conforter les plans communaux de sauvegarde et valoriser l'engagement et le volontariat lors de l'examen de la loi ma. retiens particulièrement la reconnaissance de la nation du sacrifice ultime des sapeurs pompiers par la création de la motion mort pour le service de la République et la reconnaissance des enfants de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires décédés en service comme étant pupilles de la République. Nous devons aujourd'hui adapter nos politiques et nos territoires en renforçant la prévention et les moyens de lutte tout en accélérant le reboisement post-incendies ce texte y contribue et insère également un volet d'optimisation de gestion de nos forêts, élément central du modèle à construire pour les années à venir, en commission mixte paritaire, nous avons affiné le texte dont je retiens 3 apport d'abord la simplification de la stratégie nationale. Qui optimisera les moyens de l'État et la conservation de l'obligation de l'élaboration d'un plan de protection des forêts contre l'incendie dans les territoires les plus les plus à risque et sa déclinaison pour chaque massifs forestiers permettant de mieux prendre en compte les spécificités de chaque territoire ensuite le travail global menée sur les obligations légales de débroussaillement une attente forte dans certains territoires qui nous apparaît aller dans le bon sens, enfin le maintien de la reconnaissance du rôle primordial des agriculteurs et la sylviculture dans la prévention des des feux de forêt à laquelle nous sommes très attachés. Le texte en l'état, permet de faire de la prévention de l'IT à la racine contre l'intensification et l'extension du risque incendie dans nos forêts mais également d'adapter nos forêts et de conforter l'aménagement du territoire comme Pierre angulaire de la protection de notre Patrimoine naturel pour l'ensemble de ces raisons le groupe Air des pires votera ce texte. Merci. Mes chers collègues, je suis particulièrement heureuse de saluer la présence dans la tribune d'honneur du Sénat d'une délégation de membres de la Chambre des députés du Mexique, conduite par le député Monsieur Roberto Lopez Garcia président du groupe interparlementaire d'amitié, Mexique, France, ils sont accompagnés par notre collègue Daniel Laurent, président du groupe d'amitié France-Mexique, pays d'Amérique centrale et président délégué pour le Mexique à travers sa visite en France, la délégation témoigne de son attachement à la dynamique des relations inter-parlementaire. Hier soir, ils se sont entretenus avec leurs homologues et plusieurs présidents de commission. La délégation doit également rencontrer différents acteurs économiques qui oeuvrent au développement de nos relations commerciales et de nos partenariats. La présence de la délégation mexicaine au sein de notre haute assemblée témoigne de la force de la relation qui qui unit le Mexique et la France et des valeurs que nous partageons. Mes chers collègues, en votre nom à tous, permettez-moi de souhaiter à nos homologues du Parlement mexicain la plus cordiale bienvenue et infructueux je souhaite aussi salut monsieur Reina. Sénateur qui est également là pour les accueillir. Merci je vous encourage. Allez salut. Nous reprenons le cours de notre discussion avec l'intervention de notre collègue Madame Laurence Harribey pour le groupe socialiste et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. 72.000 hectares ont brûlé en France en 2022, dont 30.000 en Gironde notamment dans le sud du département. Ou deux d'entre nous aujourd'hui réside. C'est la traduction d'abord de l'extension géographique du risque incendie, conséquence directe du réchauffement climatique en 2050 près de 50% des landes et forêts métropolitaine pourraient être concernés par un risque incendie élevé contre un tiers en 2010 mais aussi traduction de l'extension temporelle du risque incendie puisque les feux hivernaux devraient se multiplier en fait aujourd'hui la saison des feux, c'est toute l'année, comme le disait le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers cette PPL initié dans le cadre d'une mission d'information avant le terrible été 2022 donc à l'époque sans-Girondins à bord a été examiné dans un contexte d'urgence aggravée par la sécheresse de ces derniers mois. Nous saluons le travail transpartisan mené au Sénat par le président de la commission spéciale avec, cette fois-ci sénateur Girondins à bord, il y a les rapporteurs qui ont su intégrer au texte nombre de remarques et d'amendements. Nos propositions ont été entendus dans leur ensemble puisqu'une quinzaine d'amendement a été adopté et plusieurs autres amendements qui n'avaient pas abouti au Sénat ont été repris à l'Assemblée nationale. Nous nous réjouissons que la commission mixte paritaire était conclusive et l'essentiel de nos apports sur des mesures stratégiques et opérationnelles a été préservé. Dans le texte final. J'en cite quelques-unes, la sécurisation du régime des servitudes établies pour les pistes DFCI qui concerne spécifiquement le massif des Landes de Gascogne où près de 42.000 kilomètres de voies DFC vie n'ont toujours pas fait l'objet de servitude. Les communes vont ainsi pouvoir bénéficier du remboursement des frais de travaux mais également des frais annexes lorsqu'elle débroussaille en lieu et place des personnes assujetties aux zoo Exonération totale de TICPE pour les véhicules des services d'incendie et de secours. Des de secours que le notre groupe porte chaque année lors de l'examen du projet de loi de finances. Reconnaissance de la pratique des coupes tactique. Qui ont permis d'apporter des réponses d'urgence, lors des feux de l'été 2022 et enfin la mise en place d'une communication spécifique aux propriétaires de terrain concernés par les eaux nous regrettons, comme l'a souligné l'ont souligné les rapporteurs et le président l'exclusion des collectivités locales notamment des communes rurales du dispositif de réduction de cotisations patronales accordées en contrepartie de la mise à disposition d'employés sapeurs-pompiers pour les services d'incendie et de secours. Nous en avons fait la démonstration cet été et nous avons dû résoudre quelques problèmes difficiles. En conclusion, au-delà du texte. Nous souhaitons rapporté rappeler que les bonnes volontés ne suffiront pas et c'est sans doute la limite de cette proposition de loi l'écueil majeur dont ce texte ne pourra pas s'affranchir concerne le manque de moyens humains et financiers visant à renforcer la prévention et la lutte contre les incendies, l'État devra prendre toute sa part dans la prévention et ne pourra pas laisser pour seul responsable les collectivités ainsi que les opérateurs locaux qui manque de moyens. Cette inquiétude semble avoir été partiellement entendu puisque monsieur le Ministre, un an après. Les incendies de Gironde. Nous avons obtenu de nouveaux moyens aériens qui sont arrivés et qui nous rassure quelque part. L'étape suivante devra être l'installation de bases permanentes dans le, sur le territoire et en particulier dans le Sud-Ouest, c'est quelque chose qui est important pour nous et. Qui sera la prochaine étape. Nous sommes sur la bonne voie, même si tout le compte n'y est pas totalement et nous voterons bien entendu cette PPL je vous remercie. Conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du l'ex-du texte élaboré par la commission mixte paritaire modifié par l'amendement du gouvernement.

Qui vote contre. Qui s'abstient. Le texte est adopté à l'unanimité. Je vais suspendre Je vais suspendre la séance quelques instants pour permettre. Oh ministres hein ou à la séquence suivante de s'installer. Merci.

La séance est reprise. Bonjour. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. La parole est à madame Alexandra Borchio-Fontimp, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Puisque nous examinons les conclusions de cette commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Madame la présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. J'ai le plaisir de me retrouver. À nouveau devant vous pour acter en tant que rapporteur la fin des travaux sur la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. C'est forte de votre soutien sans faille riche de nos débats que j'ai défendu lors de la commission mixte paritaire les apports du Sénat auprès de nos collègues députés une CMP qui s'est avérée conclusive et se. Par un vote à l'unanimité conforme au texte du Sénat. Nul doute que lorsqu'il s'agit de protéger nos enfants. Le consensus s'impose le bon sens et l'intérêt des mineurs ont chassé les postures politiques ainsi, nous pouvons tous nous féliciter que nos deux assemblées soit parvenus rapidement à un accord sur un sujet ô combien fondamentale qu'est la protection de nos enfants. Avant de poursuivre, je tiens à vous remercier pour votre engagement pour votre confiance tout au long de mes travaux. Bien évidemment. Permettez-moi d'abord, une pensée particulière à mes collègues de la commission éducation sous la présidence bienveillante de Laurent Lafon et l'oeil avisé de Max Brisson. Cette proposition de loi, hé bien c'est le fruit d'un constat alarmant Internet peut tuer les réseaux sociaux peuvent tuer et je continuerai à dire et écrire que le harcèlement est un fléau qui gangrène nos plus fragile depuis bien trop longtemps et qu'il est temps de porter haut et fort des politiques publiques visant à protéger les victimes, celles qui dans les couloirs d'un établissement scolaire ou en parcourant parcourant ligne d'un message et ne sur les réseaux qui deviennent d'ailleurs antisociaux plonge celui qui reçoit ces invectives dans une spirale infernale. Très loin d'être un espace préservé des violences la sphère internet accentue la cruauté parce que désormais, celui qui accuse attaque critiques insultes porte un masque un masque offerts par les réseaux sociaux qui autorise l'anonymat permettant ainsi au harceleur de déverser leur haine en toute impunité diffamation calomnie agressivité aucun garde-fou ne les arrête et vous connaissez tous ici combien le harcèlement peut. Anéantir la vie des adolescents. Pour autant, nous ne pouvons pas adopté une posture qui ne serait ni comprise ni adapté que nous le voulions ou non ces réseaux font maintenant partie de notre vie. Les tablettes remplacent peu appeler chez les chercheurs en optique ne cesse de rendent les vers de plus en plus innovants pour s'adapter à la sur-, utilisation des écrans et les prescriptions des ophtalmo épuise les stocks de larmes artificielles. Internet et ses réseaux sociaux dont la diversité de cesse de nous étonner font partie intégrante du quotidien de la génération Z, rendez vous compte. Mes chers collègues né dès la naissance de nos enfants, certaines plateformes leur crée automatiquement une identité numérique. Une double vie réelle et fictive s'installent chaque jour et nos enfants n'ont pas toujours les armes pour affronter la réalité du virtuel. Bannir les réseaux sociaux reviendrait à nier l'époque dans laquelle ils vivent et serait le simple aveu de notre défaillance à les comprendre, pour mieux les adapter. La proposition de loi sur laquelle nous allons nous exprimer une dernière fois n'a pas pour objet de priver les jeunes de l'accès à un réseau social, mais bien d'adapter une réponse. D'apporter une réponse adaptée aux abus née d'un usage précoce et non encadrés. Je vous rappelle que la première inscription sur un réseau social intervient vers huit ans et demi et la plupart du temps sans que les parents en soient informés. Cette proposition de loi par de cette réalité loin d'exclure d'Internet touts les mineurs le texte à la volonté farouche de protéger les plus jeunes en créant une véritable majorité numérique en dessous de 15 ans, l'inscription à un réseau social se fera dorénavant avec l'autorisation parentale au-dessus de cet âge qui coïncide avec l'entrée au lycée le mineur pourra s'y inscrire librement au cours de nos travaux et de mes réflexions. Il m'est apparu donc essentiel de remettre au coeur de ce texte, l'autorité parental. Par facilité ou par faiblesse. Nous avons trop tendance à imputer les vices d'Internet et de ses réseaux co-, créateur des contenus diffusés et même parfois à cette heure du tout numérique en tant que parlementaire, mais on veut tout en en tant que mère de famille. Permettez-moi de vous dire mes chers collègues, que nous nous leurrons les parents aussi bien sûr porte la responsabilité d'usage que font leur enfants d'Internet. Bien souvent dépassés par une jeunesse qui ne comprennent plus et par l'évolution trop rapide de la technologie. Ils préfèrent abandonner alors à ses parents je veux leur dire ce matin de ne pas baisser les bras. La meilleure protection que vous pourrez offrir à vos enfants, hé bien c'est vous enfin avant de conclure, je voudrais me tourner maintenant vers l'avenir à court terme, il nous faudra être particulièrement attentif. Quant à l'application des dispositions de cette future loi et nous comptons sur vous Madame la Ministre et Monsieur le Ministre pour rappeler aux plateformes leurs nouvelles obligations et puis nous débattrons dès la semaine prochaine sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique sur lequel le Sénat a réuni une commission spéciale cette proposition de loi, en tout cas j'en suis convaincu, en constitue la première Pierre. Et c'est pour cette raison, et au nom de la protection de nos enfants que je vous propose d'adopter le texte issu des travaux de cette CMP. Je vous remercie. Merci madame la rapporteure. Je. C'est de la parole à présent à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Madame la présidente, madame la Ministre, Monsieur le président de la commission, madame la rapporteure mesdames et messieurs les sénateurs, nous voici arrivés au terme du parcours législatif de ce texte qui fera date et je veux féliciter madame la rapporteure pour les travaux qui en commission, puis en séance publique puis en CMP ont permis en quelques mois l'adoption de ce texte car nos enfants ne pouvait plus attendre car nos enfants sont. Les principales victimes des travers de la société numérique. Vous l'avez rappelé madame la rapporteure. Surexposition aux écrans addiction aux réseaux sociaux cyber harcèlement Exposition précoce à des contenus inappropriés autant d'atteintes brutale à leur innocence. Autant de violence psychologique faite à une génération. Qui risque bien d'être. Sacrifiée si rien n'est fait. C'est la raison pour laquelle il faut agir et c'est la raison pour laquelle la France depuis quelques années, a agi. Et a montré la voie. Au niveau national avec un certain nombres d'initiatives certaines d'origine parlementaire sur le contrôle parental sur le cyber harcèlement scolaire. Au niveau international avec des initiatives multipartite comme l'appel de Paris et le Forum de Paris pour la paix. Avec des initiatives européennes et et j'y reviendrai, mais également avec des initiatives qui ne passe pas nécessairement par la loi. Et je pense en particulier à l'engagement du ministère de l'éducation nationale et et le ministère de l'Économie et des Finances qui ont permis que à la rentrée prochaine tous les élèves de 6ème bénéficie d'un passeport numérique qui les sensibilisera aux risques et aux gestes à adopter lorsqu'ils sont victimes ou témoins de cyber-, harcèlement. Je pense également à l'engagement de madame la secrétaire d'État chargé de l'enfance et du ministre des solidarités pour qu'avec le site je protège mon enfant Point gouv Point FR tous les parents de France puisse se tourner vers une plateforme où ils pourront trouver. Des éléments susceptibles de les accompagner dans la parentalité numérique, c'est-à-dire dans la manière dont ils peuvent accompagner leurs enfants. Dans l'espace numérique et avec Charlotte Caubel, nous avons lancé il y a quelques mois une campagne nationale de communication sur cette plateforme d'outils à disposition des parents, puis je le disais, la France a agit au niveau européen en portant là l'année dernière lorsqu'elle présidait l'Union européenne un règlement sur les services numériques, un règlement majeur qui fait entrer les grandes plateformes dans l'air de la responsabilité en leur imposant un certain nombre d'obligations d'interdiction d'ordre général. L'obligation de modérer les contenus illicites sur leurs plateformes de faire auditer leurs algorithmes, par des autorités. De partager leurs données avec les chercheurs de manière à ce que puisse être identifié identifié et qualifié les dérives que nous dénonçons aujourd'hui mais aussi des obligations et des interdictions, qui vise la protection de l'enfance en ligne je pense à l'obligation qui leur est faite de publier les conditions générales d'utilisation de manière facilement compréhensible par des enfants. Je pense à la l'obligation qui leur est faite d'assurer le plus haut niveau de sécurité, de sûreté et de protection de la vie privée pour les enfants et à l'interdiction qui leur est faite. De faire de la publicité ciblée sur les mineurs. Autant d'obligations et d'interdictions qui seront sanctionnés par des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Voir. Jusqu'au bannissement. En cas de manquement répété. Nous avons agi, mais il nous faut aller plus loin, aller plus loin avec le projet de loi qui vise à sécuriser et réguler l'espace numérique a été examiné en commission spéciale. Avant-hier au Sénat et qui sera examiné la semaine prochaine en séance publique qui tire les leçons d'un certain nombre de travaux et notamment de travaux sénatoriaux sur l'Exposition des mineurs à la pornographie et je salue la contribution à ces travaux de madame la rapporteure notamment mais aussi des travaux du Sénat portant sur. La souveraineté numérique et l'équité commerciale sur le marché de l'informatique. l'informatique. En nuage aller plus loin avec ce texte que nous dont nous examinons la la version de la CMP aujourd'hui ce texte qui vise. À faire en sorte que désormais. Les grandes plateformes de réseaux sociaux vérifie l'âge de leurs utilisateurs. Et lorsque ses utilisateurs en moins de 15 ans qu'ils recueillent le consentement parental. C'est un texte fondamental car s'agissant de la protection des mineurs en ligne. La mère des batailles, c'est bien la vérification de l'âge, je constate qu'après avoir été adopté à la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale. Puis à l'unanimité au Sénat, le texte de la CMP a été adopté, lui aussi, à l'unanimité, c'est la démonstration éclatante, s'il en était besoin, que lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant est en jeu. Le Parlement s'est trouver les voies du consensus. Pour la suite. Soyez assurée, madame la rapporteure mesdames et messieurs les sénateurs qu'avec. Madame la Ministre chargé de de l'enfance, nous veillerons à ce que ce texte puisse appliquer dans les meilleurs délais, de manière à ce que. Nos enfants soient mieux protégés et d'ici là je vous invite évidemment à soutenir ce texte, que le soutien le que le gouvernement soutient également, je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre, j'invite à présent madame Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargée de l'enfance à prendre la parole. Madame la présidente. Monsieur le ministre, madame la rapporteure. Monsieur le président de la commission mesdames et messieurs les sénateurs. Je suis très heureuse d'être présent avec vous aujourd'hui pour examiner définitivement ce texte porté par le président Marcangeli après plus de 6 mois de travail efficace entre le Sénat et l'Assemblée. Très heureuse d'être présente aujourd'hui pour adresser un message clair aux enfants, aux parents et aux plateformes oui internet est un espace de liberté de découvert d'éducation d'émancipation mais il est aussi le lieu de menaces multiple qui pèsent plus particulièrement sur les enfants. Vous les avez toutes décrivent. Je ne vais pas rentrer dedans mais vraiment je crois qu'aujourd'hui tout le monde en a conscience. Ce texte porte aujourd'hui une conviction partagée avant 15 ans, les enfants sont trop jeunes pour évoluer seul dans l'espace numérique. Pour moi, cette proposition de loi nous propose un outil supplémentaire pour agir efficacement et protéger nos enfants, face aux risques que peut représenter le numérique. Elle est une Pierre dans notre mobilisation collective Capel cette révolution numérique que nous vivons maintenant au quotidien. Cette mobilisation, vous l'avez compris dans les propos de Jean-Noël Barrot. Le gouvernement est pleinement dedans à l'occasion du comité interministériel de l'enfance ou la Première ministre a fixé comme priorité une des 5 priorités, la lutte contre la la et les dangers du numérique pour les enfants. dans la suite de l'impulsion donnée par le président de la République, ce qui fait que depuis avec Jean-Noël Barrot nous travaillons sans relâche avec les plateformes pour renforcer leur responsabilité les inciter à réguler les contenus inadaptés à retirer les contenus illicites et protéger toujours et encore les enfants. Le ministre est revenu sur les réponses très concrètes qui sont apportées dans le projet de loi numérique qui est actuellement en discussion au sein de votre haute assemblée. Cette mobilisation, c'est la vôtre aussi au Sénat et vous le démontrer encore aujourd'hui avec les débats constructifs est éminemment consensuelle que vous avez eu autour de ce texte. Je tiens à saluer le travail que vous avez mené madame la rapporteure pour aboutir à cet accord entre les deux chambres. Mais ce combat, nous ne pouvons pas le mener seuls, nous devons l'affronter ensemble mais aussi avec les parents, nous ne pourrons pas gagner ce combat sans jeu aujourd'hui ils sont perdus, ils sont inquiets. Cette inquiétude fait écho au drame récent que nous avons connu et beaucoup de parents se demandent comment élever leurs enfants sereinement quand Lucas Dina l'Insee et malheureusement tant d'autres se sont donnés la mort parce que leur vie était devenue insupportable à cause du harcèlement scolaire et du cyber harcèlement de notion d'ailleurs qu'il ne faut plus séparé tant elles sont éminemment. Il n'y a que du harcèlement. Le harcèlement existe à l'école, c'est vrai et le ministre de l'éducation nationale est pleinement mobilisée pour enrayer ce fléau. Mais plus largement pour éduquer les enfants à une pratique sécurisée et du numérique. Cependant, les réseaux sociaux ont donné un nouvel écho à cette violence. Vous l'avez dit madame la rapporteure, insultes, menaces, moqueries tous ces contenus reste en ligne désormais et ne laissent aucun répit aux victimes de harcèlement. Mais au-delà de ce fléau qui nous touche profondément, on le voit entre nous mais aussi avec les enfants, le téléphone est omniprésent dans les familles le numérique et l'appareil sont au coeur de la parentalité. C'est d'ailleurs pour cette raison que Bruno Studer a très logiquement choisit de rattacher le numérique à l'exercice de l'autorité parentale. Pour ma part, j'aime bien parler de responsabilité parentale. Grâce au présent texte au-delà du principe posé par Monsieur Studer nous complétons le dispositif avec un repère très clair pour les parents et les enfants de moins de 15 ans car les parents doivent être accompagnées avec des outils et des repères très clair, ce sont évidemment, par exemple, les ateliers de la parentalité numérique comme parents parlons. Que nous avons lancé mardi dernier avec Meta pour donner aux familles des repères et des outils qui leur permettent de mieux appréhender les comportements et les usages du numérique de leurs enfants, c'est aussi le texte que vous aviez adopté sur le contrôle parental par défaut. Pour conclure Mesdames et messieurs les sénateurs, ce texte que je soutiens, est une nouvelle étape qui traduit notre mobilisation collective, pour protéger les enfants, avec des outils concrets pour y arriver. Mais il doit aussi envoyer un signal clair et créer trois dynamiques différentes une dynamique au sein des familles pour ouvrir un dialogue entre les parents et les enfants, vous le savez 8 parents sur 10 ne savent pas ce que les enfants font sur Internet alors même qu'ils vont poser des questions dans le réel ou vous allez où vous sortez qui vous voyez jamais cette question déposée sur Internet. Une dynamique à l'école et dans tous les lieux d'accueil d'enfants avec une logique de prévention et d'équité territoriale, et là on retrouve une un investissement très fort bien évidemment du ministre de l'Éducation nationale mais aussi des collectivités territoriales et plus largement une dynamique collective et sociétal. cette révolution numérique doit nous donner l'occasion de nous interroger sur nos pratiques en tant qu'adulte sur celle de nos enfants qui non on l'a dit, pas les armes pour affronter le monde numérique. Nous devons être des exemples, les accompagner et les protéger. Je vous remercie. Merci, madame la Ministre. Je rappelle qu'en application de l'article 42 alinéa 12 du règlement, le Sénat statut par un seul vote sur l'ensemble du texte. Nous passons aux explications de vote, des groupes à raison d'un orateur par groupe. La parole est donnée à madame Annick Billon, madame la présidente. Du groupe. Union centriste pour cinq minutes. Madame la présidente Madame Monsieur le Ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, je tiens à remercier et féliciter la rapporteure Alexandra Borchio-Fontimp pour son travail qui a permis d'aboutir à un texte commun avec l'Assemblée nationale en 3 mois, nous avons examiné 3 textes portant protection des mineurs dans l'espace numérique. La proposition de loi devenu loi visant à lutter contre les dérive des influenceurs sur les réseaux. La proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants et enfin la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique dont il est question aujourd'hui. Cette multiplication de textes de loi visant à protéger les plus jeunes sur l'Internet illustre bien l'urgence à s'emparer du sujet. 80% des 10 1400. Consultant l'internet sans leurs parents. La proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique poursuit 2 objectifs la régulation de l'accès des mineurs aux réseaux sociaux d'une part et la lutte contre la haine en ligne. D'autre part en commission les dispositifs proposés par la sur l'Assemblée nationale ont été simplifiées 2 amendements adoptés en séance ont permis de renforcer les mesures de prévention via l'information et le contrôle du temps d'utilisation des réseaux sociaux, ces dispositifs sont des composantes essentielles de l'éducation au numérique. Je me réjouis de ces avancées, toutefois l'application effective des dispositifs et voter est loin d'être acquise. Le contrôle de l'âge des utilisateurs et mis en échec par les difficultés techniques auxquelles nous sommes confrontés. Pourtant grâce à l'initiative de Marie Mercier, la loi oblige depuis 2020 les plateformes à empêcher l'accès des mineurs aux sites pornographiques et nous devons donc tout mettre en oeuvre pour qu'elle soit enfin appliquée et que les sites qui ne s'y conforment pas soient pénalisés. Il n'est pas acceptable de laisser ses contenus majoritairement violent qui véhicule une image dégradée des femmes qu'soit accessible avec un simple clic. J'ai 18 ans, la pornographie et ses conséquences doivent se conformer à la loi. L'éducation à les sexualités souvent inexistantes ne doit pas être remplacé par ces visionnages lors des débats avec ma collègue Catherine Morin-Desailly. Nous avions présenté un amendement complémentaires obliger les boutiques d'applications logicielles à bloquer le téléchargement des applications pour lesquelles les mineurs non pas l'âge requis. Monsieur le Ministre, vous, vous vous étiez engagé à le faire aboutir dans la perspective du projet de loi sur l'espace numérique qui numérique et nous vous en remercions. Suite au travail de coconstruction menée avec la rapporteure Alexandra Borchio-Fontimp nous le représenterons dans les jours à venir. Les précédentes lois ont permis de déployer un bouclier ayant pour but de préserver les mineurs des dangers de l'Internet que nous savons nombreux. Nous devons donc sécuriser les dispositifs existants. Nous resterons donc aussi vigilants sur l'application du décret devant préciser les contours du dispositif de la loi Studer concernant l'établissement des listes noires et blanches de site Internet ou encore d'application l'existence aussi de profils d'âge ainsi que le filtrage des données personnelles pouvant être envoyés par l'enfant à un tiers. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe Union centriste votera en faveur des conclusions de la CMP. Ce texte est un nouveau pas nécessaire qui appelle d'autres évolutions, nous aurons l'occasion d'en reparler dès mardi dès mardi prochain à l'occasion de l'examen du projet de loi sur l'espace numérique en séance. Ce texte est donc véritablement une étape nécessaire bienvenue utile et qui en appelle d'autres. Je vous remercie. Merci madame la présidente, je passe la parole à présent à un autre collègue sénateur Monsieur Bernard Phia l'air du groupe RDSE pour cinq minutes chers. Madame la présidente. Madame et monsieur les ministres, madame la rapporteur, monsieur le président de la commission, chers collègues. D'autre groupe RDSE se satisfait que la CMP sur la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne soit conclusive. Si personnel je m'en réjouis comme élus mais aussi comme médecin et comme parent. Réjouis que le législateur est pu fixer un âge. Témoin de maturité suffisante à partir duquel un mineur sera reconnu comme aptes à s'inscrire, seul sur un réseau social. Me réjouit aussi que nous ayons pu entende la voix de ses enfants isolés en souffrance à la fois dépassé apeurés et attirés par les écrans. Réjouit également que les parents puissent être pleinement. Dans la relation qui lie le mineur et les outils numériques. Et réjoui enfin que l'Assemblée nationale et le Sénat et su dépasser les postures partisanes pour s'unir autour d'un projet commun, celui de protéger nos enfants. Ensemble nous avons admis que les réseaux sociaux pouvaient être à la fois un lieu de rencontres et de solitude de culture et de désinformation de bienveillance et de haine d'opportunité et de danger. Ensemble, nous avons pris nos responsabilités face au fléau de l'addiction de la dépression et du cyber harcèlement. Afin que cette loi puisse s'appliquer le plus vite et le plus facilement possible nos deux à Lens. Ont su faire preuve d'adaptation et de simplification. Une adaptation aux familles monoparentales, notamment en précisant que l'autorisation d'un seul parent sera suffisante pour l'inscription sur un réseau social. Une simplification aussi en supprimant les réseaux sociaux labellisé, lesquels sont apparus complexe et long à mettre en oeuvre. Je salue également la mobilisation conjointe de l'Arcom et de la CNIL. Et la qualité de leur expertise mise au service de la protection de nos libertés. Ce travail en commun sera une préparation utile au moment où nous nous apprêtons à débattre du projet de loi visant à sécuriser et à régulariser réguler l'espace numérique. Toutefois. Et alors que l'actualité rend tristement compte du besoin d'agir en matière de harcèlement d'agir rapidement. Je regrette que le rapprochement entre les plateformes téléphoniques, 30, 18 et 30 20 n'est pas au fait l'objet d'une attention plus approfondie. Néanmoins cette loi s'inscrit dans un contexte où la préoccupation de la régulation numérique et croissante à l'échelle nationale comme européenne. La validation de la Commission européenne permettra d'une part de veiller à la conformité au droit de l'Union européenne et d'autre part de donner toute la force juridique nécessaire à un texte concret humain et protecteur. Le groupe RDSE votera bien entendu en faveur de ce texte. Merci. Merci. Si cher collègue, la parole est à présent à Madame Toine bourrin du groupe les républicains. Vous avez 5 minutes, chers collègues.

Madame la présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Monsieur le président de la commission, madame la rapporteure. Mes chers collègues. La commission mixte paritaire a pu parvenir sans difficulté à un accord sur les dispositions restant à débattre entre les 2 assemblées. Ainsi, hormis quelques modifications d'ordre rédactionnel, c'est le texte issu des travaux du Sénat qui a été adopté. Les améliorations apportées au texte par notre Haute assemblée vice-principalement la procédure de reconnaissance de la majorité numérique à 15 ans de l'article de mais elles introduisent également de la pédagogie avec des mesures renforçant la prise de conscience pour les enfants comme les parents des dangers d'Internet. Tout d'abord sur la majorité numérique, le Sénat a tenu à ce que le message par la proposition de loi soit clair. Aucun n'enfant de moins de 15 ans ne doit pouvoir s'inscrire sur un réseau social sans accord parental. Je suis intervenu pour une parfaite application de ce principe lors de la commission mixte paritaire pour éviter la réintroduction d'une disposition adoptée par l'Assemblée nationale puis supprimée par le Sénat qui proposait la création d'un Label pour des réseaux jugés consultable par des moins de 13 ans. On peut comprendre la volonté de distinguer les réseaux sociaux, selon leur nature mais une telle labellisation semble aussi complexes que risqués en effet. Quels seraient les critères retenus. Quelle serait l'autorité octroyant ce Label. De plus, le message véhiculé par la proposition de loi se trouverait brouiller. Ainsi que je l'ai expliqué en commission la majorité numérique comme la majorité civique ne doit pas varier selon les critères changeants. Une règle doit toujours être de portée générale, si nous voulons conserver l'universalité de la loi qui plus est dans le domaine du numérique. Je me réjouis donc que les députés nous est suivi sur cette voie. Nous avons d'ailleurs pris en considération la nature de certains sites internet en excluant notamment du Champ d'application de l'article de les encyclopédies en ligne et les répertoires scientifique à but éducatif comme le site Wikipédia afin de ne pas restreindre leur fréquentation. Autre point notre rapporteur a fait preuve de pragmatisme en proposant que l'accord d'un seul parent soit suffisant pour accepter l'inscription d'un mineur de 15 ans sur un réseau social. Un seul parent pourra également s'y opposer. Cette disposition est cohérente avec le droit existant car l'accord des deux parents est en général, réservé aux événements les plus importants de la vie du mineur comme une intervention chirurgicale ou un changement d'école et non aux actes de la vie courante mais surtout la procédure s'en trouve accéléré et simplifié et un éditeur de contenu ne pourra pas se retrancher derrière la difficulté à recueillir l'accord des deux parents. Dans le cas par exemple de parents séparés. Le travail de notre rapporteure dont je tiens à saluer l'investissement et l'écoute a permis d'apporter ces précisions. Elle s'est également montrée vigilante pour que l'on ne puisse accuser le dispositif mis en place, de contrevenir aux libertés individuelles. Le texte prévoit ainsi que la Commission nationale de l'informatique et liberté, la CNIL sera garante du respect des données personnelles, elle rendra un avis sur le projet de décret qui fixera les mots, les modalités d'application du dispositif de protection des mineurs de 15 ans. Enfin, comme je l'ai indiqué au début de mon intervention, je souhaiterais souligner l'importance de de mesures visant l'amélioration de l'information des mineurs qui s'imposeront aux entreprises de réseaux sociaux. D'une part celles-ci auront l'obligation d'informer l'utilisateur de moins de 15 ans et l'utilisateur de l'autorité parentale lors de l'inscription sur les risques liés à l'utilisation d'Internet ainsi que sur les conditions d'utilisation des données. En effet, si certains opérateurs ont déjà mis en place cette éducation aux usages numériques. Elle est loin d'être généralisée d'autre part, chaque parent a pu constater que l'enfant ou l'adolescent plongé dans son écran père sensiblement la notion du temps et n'est finalement pas conscients des heures qu'ils consacrent aux réseaux sociaux et à Internet. Dorénavant, les entreprises de réseaux sociaux auront l'obligation d'activer un dispositif de contrôle du temps passé devant l'écran et devront envoyer des notifications régulières. Prendre conscience du temps passé sur un réseau social est un 1er pas pour lutter contre l'addiction à ces plateformes. Car la meilleure défense pour les jeunes seraient qu'elles viennent de même de la compréhension qu'ils peuvent avoir, d'être finalement le jouet des réseaux sociaux. Je terminerai mon propos en saluant l'initiative parlementaire qui a permis l'élaboration du présent texte, certes, cette proposition de loi n'est qu'une étape et nous sommes conscients des difficultés techniques qui vont ralentir sa mise en oeuvre mais nous aurons fixé les bases d'un nouveau cadre de responsabilisation des plateformes et des réseaux sociaux. Ce qui est capital pour protéger nos jeunes qui on le veuille ou non sont appelés à vivre avec ces outils. Je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Claude a duré. Monsieur le président du groupe des indépendants et vous avez 5 minutes, président. Madame la présidente madame et monsieur les ministres, madame la rapporteure, mes chers collègues. Les réseaux sociaux sont devenus l'une des principales menaces contre nos démocraties. Disait il y a peu. Barack Obama dans des Atlantique. Cette phrase peut paraître grandiloquente. Elle ne l'est pas. Le rêve de quelques Guy californien du début des années 2000, d'un Internet, porteur d'une connaissance universelle d'une transparence inédite. Et de nouveaux Liens sociaux à l'échelle de la planète s'est transformé en une réalité beaucoup plus prosaïque avec News. Discours de haine harcèlement désinformation manipulation électorale à grande échelle ferme eux à trolls ne sont que quelques exemples des dérapages d'une technologie qui connaît un succès mondial, mais bien souvent, pour de mauvaises raisons. Ces dérapages. Tout le monde en est victime. Mais certains sont plus victimes que d'autres. Il s'agit des adolescents dont la personnalité est en construction et qui sont mal armés pour résister à ces risques adolescent n'est en fait pas le terme adéquate puisque nous savons que l'âge moyen de primo-. Inscription à un réseau social intervient désormais vers l'âge de 8 ans et demi, vous ne l'avez rappelé madame la rapporteure. La plupart du temps, avec un contrôle parental minimum voire absent. Depuis peu un nouveau venu a rejoint, Facebook, Twitter, Instagram et quelques autres. Leurs algorithmes était addictif le sien entraîne une véritable dépendance et bien entendu, tous se sont empressés de suivre dans cette course à l'échalote de la su études ou la qualité des contenus et l'intérêt des enfants a été jetée depuis bien longtemps par dessus bord au profit de la seule chose qui compte les heures passées devant l'écran qui garantissent des espaces publicitaires maximum donc des profits maximum. Voilà qui est l'Internet des années 20, telle que nous la montré la commission d'enquête sur TikTok dont nous allons rendre les commissions, les conclusions dans quelques jours. Le texte que nous examinons aujourd'hui je voudrais en remercier Laurent Marcangeli. Ce texte était nécessaire. Il ne sera suffisant que s'il est réellement mis en oeuvre. Après des années d'insouciance. Nous commençons à nous réveiller. Le RGPD puis le DSA et le DMA sont aujourd'hui les témoins de cette prise de conscience. Ils ne seront efficaces que si elles sont appliquées. Faire une loi et ne pas la faire appliquer cette autorisé ce que l'on veut interdire disait Richelieu. Le législateur aujourd'hui il fait son travail. En tout cas, il entreprend cette aux exécutifs que revient désormais la responsabilité de l'action. Je suis un Européen convaincu mais je vous le dis, Monsieur le midi je vous l'ai dit la semaine dernière lorsque nous nous sommes rencontrés le dans la commission d'enquête. Si l'application de ces textes européens devait être confiée à des organismes insuffisamment doté. Si les remontées prévu de toutes les infractions au niveau européen devait prendre des années comme cela commence à être le cas avec la diffici Si les voies de recours, on devait prendre des années supplémentaires. Si chaque pays n'avaient plus la possibilité de sanctionner les principales infractions commises sur son territoire. Alors les Gafam et les autres après, une fois de plus gagné la bataille de retardement qu'il mène depuis des années avec leurs années leurs armées de lobbies c'est de juristes avec leurs milliards qui leur permettent de traiter par l'indifférence. Les amendes qui leur sont infligés dérisoire pour eux même lorsqu'elles sont significatives, elles sont désormais inscrites dans leurs comptes au titre des provisions pour imprévus. La main des gouvernements démocratiques ne doit plus tremblé. Monsieur le Ministre Madame la Ministre et vous laisserez votre nom dans la fonction que vous exercez. Si vous y parvenez. Vous avez vu tout à l'heure des paroles fortes et je vous en félicite. Mais c'est sur les actes que vous serez jugé je le dis avec force si les mesures de contrôle de l'âge des utilisateurs des applications ne sont pas strictes. Si le contrôle par les États de la mise en place de mécanismes de surveillance réellement efficace par les plateformes n'est pas réalisé et la menace de l'interdiction clairement exprimée. Et si, par conséquent, les enfants de 8 ans comme les adolescents, continuent à voir leur attention la construction de leur psychisme et la réussite de leurs études compromise par des entreprises d'abrutissement et pour utiliser le terme d'un chercheur de crétinisme digital. Alors nous aurons perdu la bataille de l'éducation de l'instruction et de l'équilibre psychologique qui est déjà depuis des années, bien mal engagée. C'est là le défi auquel s'attèle aujourd'hui le Parlement c'est la votre défi madame et monsieur les ministres, et c'est en définitive comme le disait Obama dans la citation du début de mon intervention, je pèse mes mots. Un des défis auxquels sont confrontées nos démocraties. Je vous remercie. Merci monsieur le président. La parole est à présent à monsieur Thomas de dessus du groupe des écologistes et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente madame la rapporteure Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans un mouvement plus large de régulation du monde numérique et particulièrement de la protection des enfants dans cet espace. Ce n'est pas la première fois que notre haute assemblée se penche sur la question. Proposition de loi visant à lutter contre le cyber-harcèlement, commission d'enquête sur TikTok, proposition de loi protégeant le droit à l'image des mineurs en ligne. Le Sénat est au rendez vous des enjeux du numérique. La spécificité de ce texte et qu'ils traitent plus particulièrement des plateformes de réseaux sociaux sur lesquels les jeunes sont particulièrement exposés à des contenus violents pornographiques. Ou illicites. La mesure phare de ce texte est une mesure de principe importante. Elle fixe là une majorité numérique à 15 ans en dessous de laquelle l'accord parental est indispensable pour l'inscription sur un réseau social. Ce texte propose également d'inscrire pour la première fois dans la loi une définition juridique des plateformes de réseaux sociaux reprenant celle du DMA européen l'obligation pour les opérateurs de réseaux sociaux de diffuser de diffuser des messages de prévention contre le harcèlement ainsi qu'un cadre plus contraignant dans lequel les opérateurs de plateforme en ligne doivent répondre aux réquisitions judiciaires. Dans le cas d'une enquête préliminaire ou de flagrance la navette parlementaire a utilement enrichi ces dispositions et celui qui nous est proposé aujourd'hui. Après la commission mixte paritaire va dans le bon sens. Toutefois malgré la qualité de ses intentions, je reste toujours dubitatif sur la mesure de contrôle d'âge via le référentiel établi. Par l'Arcom. Qu'est-ce qui nous est proposé ici une responsabilité donnée aux plateformes de s'assurer qu'aucun enfant de moins de 15 ans, on accède aux réseaux sociaux sans l'autoroute sans le. L'autorité de leurs parents en se conformant un référentiel établi par l'Arcom après avis de la CNIL. On parle ici du même référentiel qui occupera une grande partie de nos débats la semaine prochaine lors de l'étude du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Le contrôle de majorité est une question. Quasi aussi vieille qu'Internet cela fait plusieurs années que l'Arcom et la CNIL se penche sur le sujet et il faut le dire les choses. Il faut dire les choses comme elles le sont, c'est-à-dire la solution technique n'existe pas à l'heure actuelle, l'équation à résoudre entre contrôle d'âge, protection de la vie privée et sécurité, donner des données paraît pour l'instant difficile à résoudre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CNIL elles-mêmes dans un rapport de 2021, je cite, s'agissant de la vérification d'âge les dispositifs existants ou envisagés sont généralement insatisfaisant à 2 titrent certains repose sur une collecte massive de données personnelles et apparaissent dès lors difficilement conforme aux principes de de propreté qui sont des données, d'autres moins intrusif sont cependant inefficace parce que trop aisément contournées par les mineurs. Ce problème n'est pas uniquement français à l'heure où je m'exprime aucun pays du monde on a réussi à trouver la solution technique efficace et respectueuse des libertés publiques pour s'assurer du contrôle là j'en ligne. À cela s'ajoute que, même si une solution robuste et française. De contrôle d'âge voient le jour. Les solutions de contournement font déjà leurs preuves. J'ai souvenir dans cet hémicycle du président du précédent chargé du numérique Monsieur Cédric O faisant en Direct ici à votre place. Monsieur le Ministre de la démonstration de son VPN pour changer virtuellement de pays, vous me direz que c'est une solution de spécialistes de connaisseurs et pourtant pourtant les vendeurs de VPN sont aujourd'hui. Depuis des années les partenaires privilégiés des jeunes vidéastes sur YouTube ce ce qui s'adresse à la jeunesse. Nous sommes là au coeur des problèmes d'une régulation nationale d'Internet. Ainsi, nous comprenons l'intention du législateur avec cette PPL et nous la trouvons louable mais force est de constater qu'il y a un risque qu'elle ne reste qu'un voeu pieux nous débattrons plus profondément du référentiel devant servir au contrôle d'âge la semaine prochaine. Toutefois, ce texte a un intérêt majeur, celui d'ouvrir le dialogue entre les femmes dans les familles sur l'accès aux plateformes pour les adolescents en fixant cet âge de majorité numérique nous fixons une limite. L'association des parents au dispositif prévu par la loi pourra faire naître un échange fertile entre les générations, une responsabilisation quant au bon usage d'Internet l'éducation, l'accompagnement des enfants dans la découverte du numérique. La pédagogie c'est un enjeu majeur de la protection des mineurs. Cette proposition de loi, il concourt. C'est pourquoi le groupe écologiste votera pour. Je vous remercie, cher collègue, la parole est à présent hein monsieur Julien Bargeton, sénateur du groupe RDPI et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame Madame la présidente madame la rapporteure Monsieur de la commission, madame et monsieur les ministres. Notre groupe se réjouit également que nous puissions aboutir à un texte à l'issue de la commission mixte paritaire sur cet important projet d'une majorité numérique. Cela fait évidemment partie. Des éléments qui sont constitutifs d'une régulation progressive du numérique. En France, ce texte comprend plusieurs éléments, ils ont été détaillées. Je n'y reviens pas. L'essentiel, ce sont bien sûr des obligations fixées aux plateformes et la principale obligation c'est de dire que il n'y a pas d'inscription avant l'âge de 15 ans sauf l'accord, l'accord d'un des 2 parents il y a ensuite évidemment une série d'autres obligations toujours la possibilité pour les parents de suspendre le compte d'un mineur si le le souhaite une série. Donc ça c'est le contrôle puis il y a une série aussi d'information d'information sur les risques en matière de cyber harcèlement le fait aussi d'inviter les usagers les utilisateurs à pouvoir signaler tous les comportements prohibés. Bref, une série de mesures qui sont utiles pour la protection des mineurs et qui évidemment répondent à un certain nombre d'enjeux qui ont été régulièrement posée par notre assemblée. Il est vrai qu'il y a eu 2 points d'attention dans ce texte. Il y a eu un débat. Sur le fait d'interdire totalement au delà. En dessous de 13 ans mais je crois que c'est important de rappeler que l'esprit de ce texte est bien celui d'accompagner la responsabilité parentale c'est-à-dire que c'est évidemment l'accompagnement des parents pour instaurer un dialogue au sein de la cellule familiale sur l'utilisation des réseaux sociaux ce qu'ils peuvent apporter mais aussi les dangers qu'ils représentent pour le mineur. Et puis aussi toujours le fait de respecter le droit européen, ce qui est évidemment extrêmement important, il ne faut pas que cette loi Vienne empiéter ce qui relève de l'échelle européenne, ça a été dit les marchés numériques comme les services numériques le DMA, d'un côté et le DSA, de l'autre et donc il la première version avait tendance à être pour partie incompatible avec la réglementation européenne. Cela étant dit, il est vrai que nous devons porter ce faire ce combat au niveau européen pour pouvoir. Imposer davantage d'obligations aux plateformes travailler avec nos partenaires pour y parvenir pour que nous puissions ensuite traduire dans les faits est réellement appliquée le cadre européen telle qu'il est déjà en cours d'être appliquées mais aussi tels qu'il continue à se construire. Parce que là, le législateur nous sommes évidemment confronté à un sujet extrêmement évolutif et où donc la loi doit constamment s'adapter aux évolutions du secteur. On pourrait prendre un peu l'image de l'hydre de Lerne hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression parfois que le numérique apporte beaucoup mais parfois c'est. L'hydre de Lerne on coupe une tête la tête repousse et on n'a jamais fini à chaque fois on doit inventer, innover, à la mesure est à la hauteur de l'innovation des acteurs eux-mêmes c'est tout l'enjeu de la législation dans ce secteur et qui est un peu nouvelle pour nous, puisque au fond les parlements auparavant légiférer plutôt pour le temps long. Il y avait un temps ont voté une loi en prenait décret d'application et puis on l'appliquait on est on évaluait et etc maintenant on est dans des secteurs qui vont extrêmement vite qui bouge très rapidement et où les législateurs doit sans cesse s'adapter, c'est évidemment un peu les enjeux et cela a été dit, c'est ce qu'on a fait déjà. Avec, notamment la régulation de l'utilisation des portables dans les établissements scolaires dès 2018 hein, c'était au tout début du précédent quinquennat la encadrement des enfants influenceurs la protection du droit à l'image. Dans la vie privée pour les pour les enfants, donc ce qui a été accompli auparavant aujourd'hui ce texte qui constitue une Pierre supplémentaire, une avancée supplémentaire avant évidemment le débat qui viendra sur le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique. Nous, nous voyons bien, donc nous n'avons pas fini. Et moi je me réjouis que sur des sujets, même s'il y a des différences parfois d'appréciation des débats politiques nous parvenions à avancer dans dans un esprit consensuel parce que c'est important que face à des acteurs qui soit très puisqu'ils forme de rechercher une forme de convergence ou de consensus dont nos assemblées pour aussi pouvoir faire levier faire du judo et avoir un rapport de force parlementaire et avec le gouvernement vis-à-vis d'acteurs qui sont très puissant donc c'est ce que nous continuons à faire ce texte il contribue évidemment après déjà des textes adoptés, ce n'est pourtant loin d'être terminée et nous aurons l'occasion dès la semaine prochaine d'avoir de nouveau ce type de débat, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à Madame. Sylvie Robert du groupe socialiste et vous avez 5 minutes.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues. Nous nous retrouvons donc pour adopter définitivement la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique à lutter contre la haine en ligne. Je suis très satisfaite qu'un accord ait été trouvé la semaine dernière en commission mixte paritaire sur la version du Sénat ce qui souligne une fois de plus la qualité du travail de la chambre haute et en particulier celui de notre rapporteur Madame Alexandra Borchio-Fontimp, qui avait adopté à l'unanimité ce texte cette proposition doit s'attaque à des sujets d'importance majeure, celui de la surexposition des enfants de plus en plus jeunes, aux réseaux sociaux qui entraîne des effets désastreux sur leur santé mentale et physique et les confronte à de nombreux phénomènes n'efface-t-elle par exemple le harcèlement ou la surinformation. Cette proposition de loi donc pour objet dans son article 1er, de donner une base légale aux réseaux sociaux en ligne puisqu'aucune définition n'était alors prévu par par la loi. par la loi. Cette définition légale vise en premier lieu à protéger les mineurs des effets néfastes de surexposition à ces réseaux et à et encadrer leur présence. Ainsi un consentement parental sera requis pour l'inscription sur les réseaux sociaux des mineurs de moins de 15 ans, âge auquel est désormais fixé la majorité numérique en vertu de l'article 2. Le consentement sera recueillie sur la base d'un référentiel mis en oeuvre par l'Arcom gage de fiabilité des conditions de vérification d'âge. Je me réjouis que le texte de la CMP et repris la version du Sénat et supprimée. Le système de labellisation des réseaux destinés aux moins de 13 ans un peu usine à gaz difficile à mettre en oeuvre et un peu peu peu réaliste au regard de la présence actuelle de très nombreux petits adolescents sur les réseaux à l'article 3 des sanctions sont prévues pour les réseaux contrevenant à cette obligation de vérification d'âge avec le cas échéant, obligation de répondre au juge dans les délais resserrés. La remise d'un rapport au Parlement pour évaluer les conséquences sur la santé des jeunes de cette surexposition justifie une entorse à la jurisprudence du Sénat sur la remise d'un rapport qu'on compte tenu de l'importance de la question. La proposition de loi que nous allons définitivement adopté aujourd'hui a été enrichi du fait de la recrudescence des faits de harcèlement avec un élargissement à l'article 1 bis de la liste d'infractions contre lesquelles les fournisseurs d'accès de services en ligne doivent lutter par des informations aux internautes et des signalements à la diffusion de contenus constitutifs d'atteinte à la vie privée à la sécurité des personnes ou constituant toutes les formes de chantage ou de harcèlement. Autre enrichissement sous la pression de l'actualité, l'obligation pour les fournisseurs d'accès et de services en ligne de publier des messages de prévention contre le harcèlement et la communication des structures d'accompagnement des personnes faisant l'objet de cyber de cyber harcèlement. À noter que ce dispositif est introduit à l'article en terre de la proposition de loi reprend l'essentiel du dispositif de l'article 4 de la PPL déposée par mon groupe sous l'impulsion de ma collègue Sabine von et qui présidait la mission sénatoriale sur le harcèlement scolaire. Je me félicite que plusieurs amendements déposés par notre groupe d'adopter, comme l'obligation pour les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne de délivrer une information à l'utilisateur sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de. Et pardon, les moyens de prévention aux mineurs de moins de 15 ans ainsi qu'à leurs parents. La délivrance d'une information à l'usine. L'utilisateur de moins de 15 ans, Claire et adaptée des conditions d'utilisation de ces données et de ses droits informatique et libertés soit son droit à l'oubli, conformément aux recommandations de la CNIL, la mise en place par les réseaux sociaux, d'un dispositif permettant de contrôler le temps d'utilisation de leurs services. Lors de l'inscription d'un mineur ou encore l'amendement identique à celui de notre rapporteur sur l'exclusion du Champ d'application du dispositif des encyclopédies en ligne et des répertoires scientifique que j'avais porté, j'approuve. Par ailleurs la suppression décidée au Sénat de l'article 5 de la PPL qu'initialement, prévoyait le rendu d'un rapport sur les possibilités de fusion des plateformes d'appel pour le harcèlement scolaire et cyber harcèlement. Il me paraît enfin opportun effectivement de maintenir les deux numéros, le 30 20 et le 30 18. Chacun des 2 organismes étant spécialisé et leurs experts apporte toujours des réponses. Notre groupe des sénateurs socialiste, écologiste et républicain approuve donc ce texte même si je dois vous avouer j'émets quelques réserves sur la pratique habilité de certains des dispositifs votés comme par exemple l'élaboration rapide de référentiels par l'Arcom pour le recueillement du consentement parental à l'inscription de mineurs qui risque de s'avérer une tâche très complexe mais où nous en parlerons aussi la semaine prochaine. Par ailleurs, comme nous l'avons souligné ce texte pourra malheureusement pas tout résoudre la haine et la violence auxquelles sont exposés les jeunes sur les réseaux sociaux ne vont malheureusement pas il y a un problème d'éducation, il vaut mieux former les enfants mieux former les parents, les enseignants face à ces gens en jeu. Autre recommandation faite en son temps par la mission sénatoriale. C'est donc en toute lucidité que notre groupe approuvera bien sûr les conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi qui vise à instaurer une majorité numérique et contre la haine en ligne je vous faire. Merci cher collègue. Et enfin, la parole est à madame Éliane Assassi. Madame la présidente du groupe communiste pour cinq minutes, chers collègues. madame la présidente. Madame et messieurs les les les ministres, mes chers collègues. Cette proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique à lutter contre la haine en ligne est une réponse à une tendance qui est en effet lourde de l'accès des plus jeunes à Internet avec une première inscription, cela a été dit à un réseau social. Qui interviendrait en moyenne vers huit ans et demi et avec plus du quart des 7 disant qu'il se rendrait régulièrement sur les réseaux sociaux. Ce texte était effectivement nécessaire. Les réseaux sociaux font partie du quotidien de nos petits enfants de nos enfants et adolescents, tandis que le risque d'addiction lié à la consommation et. Réfléchie méticuleusement organisée par des multinationales mercantile. De plus, le risque de cyber harcèlement est réel. Selon une étude datant de novembre 2022 près de 60% des enfants et adolescents déclarent avoir déjà été victimes de cyber harcèlement cela vous le savez peut laisser des séquelles conduire à la dépression voire à des conduites suicidaires lorsqu'on sait que le suicide représente 16% des décès chez les plus jeunes et cas d'enfants cyber harcelé sur 2 a déjà pensé au suicide. Il est clair que nous sommes face à un enjeu national de santé publique aujourd'hui il existe un gouffre entre les obligations réglementaires des plateformes et la réalité pratique sur le terrain, en effet, alors même qu'il existe un âge minimum requis pour s'inscrire sur les réseaux sociaux. C'est plus de la moitié des enfants de 13 ans qui sont déjà inscrits sur un réseau social. À cela s'ajoute une précocité croissante dans l'accès aux smartphones exposants également de fait les les enfants aux dérives de cette technologie. Comme nous avions eu l'occasion de le dire lors de des débats ici au Sénat, nous pensons que la responsabilité des entreprises propriétaires des réseaux sociaux apparaît clairement et qu'il serait temps de les encadrer plus fermement pour qu'il respecte les dispositions qui les concernent. À cet égard, nous considérons que ni le texte au Sénat, ni la conclusion de la commission mixte paritaire de répondre convenablement à cette question. Et notamment s'agissant de la sanction. En effet, celle-ci n'est pas celle la sanction n'est pas en adéquation avec le poids économique de ces grandes entreprises et il s'agit d'un manque notable de cette proposition de loi puisque, à l'origine, ces auteurs prévoyez une amende d'un montant maximum d'un pour 100 du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. Par ailleurs, il est également prévu de faciliter les demandes d'information auprès des plateformes dans le cas d'une réquisition judiciaire dans un délai de 8h pour les cas urgents et de 10 jours pour les autres cas afin de livrer toute information utile dans le cadre d'une d'une enquête. Nous aurions pourtant préféré un délai de 48 heures pour les autres cas, comme cela avait été décidé à l'origine par les auteurs de cette loi au regard des possibles conséquences gravissimes que peuvent engendrer la lenteur des procédures enfin nous souscrivons pleinement à la demande de rapport inscrit à l'article 4 de cette proposition de loi puisque celui-ci nous permettra de gagner en efficacité par un apport de connaissances sur les conséquences de l'utilisation des réseaux sociaux sur les jeunes. Alors nous avons des points de vigilance. Nous avons des remarques mais nous considérons que cette proposition de loi constitue une première étape intéressante dans un contrôle à l'accès d'Internet pour nos plus jeunes et c'est donc dans cet esprit que mon groupe votera favorablement pour ce texte. Merci madame la présidente. Conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Qui vote pour. pour. Abstentions, félicitations. C'est une proposition de loi définitivement adoptée. À l'unanimité. Merci beaucoup. Je vais suspendre. La séance pour quelques instants afin de permettre à chacun de s'installer pour le prochain point de l'ordre du jour, la séance est suspendue.

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse. La parole est à monsieur Martin lévrier rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues. La commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse est parvenu à un texte commun lors de sa, de sa réunion le 1er juin dernier. Cette issue était attendue, tant les divergences qui opposent et nos deux chambres étaient minimes et peu nombreuses. Il convient toutefois de la saluer et de se féliciter du dialogue constructif qui a permis dans un esprit transpartisan dont Richard. La proposition de loi à chaque étape de son cheminement démocratique et j'en profite pour saluer la présence dans nos tribunes de Madame. La députée Sandrine Josso, à l'initiative de ce texte. L'accord trouvé en CMP se rapproche grandement de la version défendue par le Sénat qui a en première lecture épuré le texte de dispositions dépourvues d'effet utile et la enrichi par différents apports consensuel. L'article 1er ah prévoit la mise en place par les agences régionales de santé et d'ici au 1er septembre 2024 de parcours spécifique associant, médecins, sages-femmes et psychologue dans la prise en charge des interruptions spontanées de grossesse. Les apports du Sénat renforçant les objectifs d'information au parcours ont été retenues par la CMP. Celle-ci n'a apporté à ces dispositions qu'une modification visant à laisser aux ARS le soin de nommer ces parcours. L'autre modification de fond adoptée par la CMP est une modification de forme. Dans l'intitulé du texte, la commission des affaires sociales du Sénat avait substitué au terme fausse couche jugé stigmatisant par les associations l'expression interruptions spontanées de grossesse consacré médicalement. Cette dernière étant toutefois méconnue du grand public et afin de rendre cette proposition de loi accessible au plus grand nombre. La commission mixte paritaire, a précisé l'intitulé du texte. On le renomme en proposition de loi visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse fausse couche. Sur l'ensemble des autres articles et sous réserve des coordination rédactionnelle et juridique et qui s'imposer la version équilibrée défendue par le Sénat a été préservé, sans modification de fond. l'article 1er bé lève le délai de carence applicable à l'indemnisation des congés maladie prix consécutivement à une interruption spontanée de grossesse non seulement pour les assurés du régime général et les agents de public mais également, comme l'a souhaité le Sénat pour les indépendante et les non-salariés agricoles. Cette mesure permettra de lutter contre un non-recours au congé regrettable pour les femmes qui en ressentent le besoin. L'article premier s'est ajoutée par le Sénat, prévoit une protection contre le licenciement de 10 semaines à l'égard des femmes confrontées à une fausse couche dites tardives après la 14ème semaine d'aménorrhée afin de renforcer leur leur protection face au risque de discriminations professionnelles qu'elles encourent et de limiter les effets de seuil. La CMP a jugé que cet article compléter utilement les le texte et la adopté dans sa rédaction issue du Sénat. L'article premier adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat permettent aux sages-femmes d'adresser à un psychologue conventionnés. Dans le cadre du dispositif mon parcours psy leurs patientes, et en cas d'interruption spontanée de grossesse leur partenaire. L'article 1er a ajouté par le Sénat, vise à étendre le Champ de un rapport déjà prévu en LFSS pour 2021 portant sur l'accessibilité de mon parcours psy afin qu'il étudie spécifiquement l'accès des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse au dispositif. La commission mixte paritaire a jugé cette évaluation nécessaire. Il a donc adopté l'article telle qu'issue du Sénat. L'article 1er bis supprimé par le Sénat faisait obligation aux professionnels de santé. Dans la prise en charge des femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse d'informer leurs patientes des possibilités de traitements comme de leur implication et de leur proposer un nouvel examen médical 4 semaines après le premier. Sa suppression a été maintenu par la CMP. L'article 1er Terre qui consistait en une demande de rapport sur l'extension de l'assurance-maternité dès les premières semaines de grossesse. Une mesure jugée peu opérationnel et inopportune par la direction de la sécurité sociale avait été supprimé par le Sénat, la commission mixte paritaire. Ah là encore maintenu cette suppression. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le texte que nous hier en. Aujourd'hui a été considérablement enrichis grâce aux travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat il portent des mesures consensuelles adapté et utile qui permettra de mieux accompagner les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse et de mieux tenir compte des effets psychologiques que peut comporter cet accident de la vie. C'est pourquoi je vous invite à donner une large majorité au texte issu de l'accord en commission mixte paritaire, je vous remercie. Merci. Si cher collègue, la parole est à présent Monsieur François Braun Ministre de la Santé et de la prévention. Madame la présidente, madame la présidente de scène. Monsieur le rapporteur. Mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour cette ultime étape d'un processus législatif qui a symboliquement été entamée le 8 mars dernier par l'examen en première lecture de ce texte, à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Les votes unanimes dans cette navette parlementaire a été jalonnée ainsi que le travail constructif qui a été menée en bonne entente avec le gouvernement dans les 2 assemblées avant que les parlementaires présents en commission mixte paritaire ne s'accordent sur un texte commun nous prouve bien une chose. Le 8 mars mais aussi 365 jours par an. Il y a certains sujets qui seront toujours nous rassembler, malgré nos différences et nos divergences politiques. Lorsqu'il s'agit de faire avancer les droits des femmes. Malgré des sensibilités diverses. Le travail parlementaire peut faire l'objet d'une coconstruction associant les deux chambres et un maximum de groupes. Je m'en réjouis, je tiens à saluer. Je suis aussi avoir d'emblée un mot chaleureux pour la députée Sandrine Josso. Présente. En tribunes qui est à l'initiative de ce texte mais également pour le sénateur Martin lévrier rapporteur au Sénat ainsi que pour tous les parlementaires qui ont été nombreux à s'investir dans ce débat important. En effet, le texte que vous allez. Je le dis, j'espère sans trop m'avancer, adopté définitivement. Dans quelques instants comporte des dispositions nécessaires juste et équilibrée. Cette proposition de loi constitue une véritable avancée pour toutes les femmes tous les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse. Tout d'abord ce texte a permis de lever un tabou encore persistant autour de ce qu'on appelle communément la fausse couche passé sous silence minimiser voire souvent banalisée l'interruption spontanée de grossesse et pourtant un événement qui nous concerne, et nous affecte tous que ce soit, directement ou bien par nos proches. Ces chiffres on peut être mentionné plusieurs fois au cours de notre travail mais il faut le rappeler encore car leur ampleur est éloquente. En France, une grossesse sur cinq est interrompue par une fausse couche. On estime qu'une femme sur 10 sera confronté à cette épreuve au cours de sa vie. C'est la première cause de consultations aux urgences gynécologiques. Une fois cela dit, on comprend combien d'interruptions spontanées de grossesse avec 200.000 femmes, leur famille, leur entourage toucher chaque année un véritable phénomène de santé publique et de société. Une ampleur qui ne doit se bornant pas nous faire oublier que la fausse couche reste avant tout un drame intime que chaque femme vit dans sa Chair et de manière très différente selon son histoire de vie. Et qui touche aussi le partenaire. C'est dans cet état d'esprit qui a présidé à l'élaboration de ce texte qui n'a jamais visé à imposer des schémas préétablis ou des parcours standardisés, au contraire, il s'agit bien ici d'ouvrir des droits. C'est-à-dire de mettre à disposition des femmes et faciliter leur accès à toutes les ressources et à tous les outils nécessaires auxquels elles pourront librement avoir recours. C'est le fil rouge de la construction de ce texte qui visait initialement à mettre en place un accompagnement psychologique adapté aux femmes traversant une interruption spontanée de grossesse par un travail commun. Vous l'avez dit d'enrichissement du texte. Nous sommes finalement parvenus à mettre sur pied un véritable dispositif cohérent de prise en charge et de suivi de ce traumatisme subi par trop de femmes. Il me semble important de souligner que ce texte, à commencer par considérer les aspects psychologiques de la fausse couche. C'est tout à fait représentatif d'un changement salutaire de mentalité dans la manière d'envisager la santé. Je parlais de briser les tabous. Celui qui existe de longue date autour du bien-être et de l'équilibre psychologique est en train de s'étioler au gré des projets des progrès que nous faisons qui nous amène à considérer la santé dans une approche plus transversale et plus globale. Bien sûr, des fausses couches, en elle-même comporte des risques et des conséquences physiques importants. Mais au-delà des répercussions physiques et du nécessaire accompagnement médical la disponibilité d'un soutien psychologique est indispensable en cas d'interruption spontanée de grossesse. Alors que la parole se libère les témoignages de femmes nous prouve combien l'arrêt brutal d'une grossesse et d'un projet de maternité est un choc d'une grande violence. Il ne faut pas en sous-estimer les conséquences le stress post-traumatique, l'anxiété, l'angoisse, la dépression qui peuvent perdurer ou se manifester parfois des mois voire des années après. Il y a aussi des questions et des remises en questions, parfois même de la culpabilité qui accompagne ce drame. Il y a finalement le deuil ce deuil périnatal si particulier dans les femmes parlent mieux que moi, quand elles décrivent leur souffrance transparente aux yeux de la société ou encore ce deuil impossible souvent solitaire et sans rituel. Le texte que nous achevons d'examiner aujourd'hui j'en suis convaincu, nous permet de prendre en compte ces différents aspects et de créer dans la loi tous les outils pour accompagner celles et ceux qui font face à la double perte que représente la perte physique de l'embryon ou du foetus et la perte symbolique de l'enfant à naître et du projet de parentalité. Premièrement pour garantir à chacune l'accessibilité de cette indispensable accompagnement psychologique. Les sages-femmes seront désormais habilités à dresser leurs patientes vers des séances d'accompagnement psychologique de mon soutien psy dans tout type de situation liées à la grossesse. Je tiens à souligner le caractère inédit de ce dispositif qui permet, je le rappelle, la prise en charge intégrale et sans avance de frais de 8 séances chez un psychologue agréé. C'est une mesure qui a déjà prouvé toute son efficacité en offrant rapidement une première réponse tout en permettant une orientation vers des soins plus spécialisé en cas d'indicateurs de gravité. Notons d'ailleurs que 71% des plus de 131.000 patients qui en ont bénéficié depuis sa mise en oeuvre sont des femmes. Dans le cas d'une fausse couche le ou la partenaire de la patiente pourra également faire l'objet d'un adressage par la sage-femme. Je tiens à souligner que cette prise en compte du conjoint est un apport parlementaire qui est tout à fait légitime et bienvenue autant pour reconnaître la souffrance propres du partenaire que son rôle de soutien auprès de sa partenaire. Cette nouvelle mission c'est aussi une valorisation, une reconnaissance importante de l'engagement des sages-femmes auprès de leurs patientes, alors que nous allons justement accompagner leur montée en compétences par une jeune une réingénierie de leur formation qui sera effective dès la rentrée 2024. Dans la lignée de la loi, Rist et de la proposition de loi Valletoux, je l'envisage comme une brique supplémentaire apportée au chantier du décloisonnement des parcours de soins et de la modernisation de notre système de santé. Aussi, en second lieu c'est justement dans cette logique de parcours de soins adaptés aux besoins de chacune que s'inscrira cette prise en charge psychologique, en effet, grâce à cette loi seront mis en place à partir du 1er septembre 2024, dans tous les territoires sous l'égide des ARS un parcours spécifiquement dédié aux victimes, aux femmes Ce parcours associera tous les professionnels médicaux les hospitaliers les libéraux bien sûr les psychologues dans le cadre d'une approche complémentaire pluri-professionnelle pour accompagner au mieux chaque situation tout en développant la formation des soignants et en améliorant l'accès à l'information et la prévention à destination des couples. Finalement, alors que nous répondons aux enjeux de la prise en charge clinique et psychologique des fausses couches, il reste encore une autre conséquence à laquelle il était urgent de s'attaquer. En plus du traumatisme physique et mentale. La fausse couche fait aussi supporter un coût financier aux femmes dans le cas où elles doivent arrêter de travailler. Je refuse cette triple peine. C'était une promesse de campagne du président de la République. La Première ministre a eu l'occasion de l'annoncer le 1er mars 2023. Nous supprimons les jours de carence en cas de fausse couche pour l'ensemble des assurés. Cette proposition de loi vient concrétiser cet engagement qui sera effectif dès que possible et au plus tard au 1er janvier de l'année prochaine. Cette levée de la carence. C'est une excellente nouvelle et une avancée concrète dont nous pouvons tous être fiers. C'est aussi une solution qui permet de prendre en compte la diversité des situations de ces femmes confrontés à un phénomène et leur permettant de préserver la confidentialité et du secret médical. Je tiens à saluer ici l'ajout de l'article premier c'est par un amendement sénatorial, qui instaure une protection contre le licenciement au bénéfice de femme confrontée à une interruption spontanée de grossesse dite tardive et qui participe à lutter contre les risques de discriminations professionnelles. Mesdames les sénatrices messieurs les les sénateurs. J'ai toujours assumé de dire notre système de santé ne s'adapte pas assez vite aux spécificités des femmes qui ont trop longtemps été marginalisées dans la prise en charge clinique comme dans la recherche. Depuis mon arrivée au ministère, j'ai fait de la lutte contre les inégalités de santé, ma priorité. Et je pense en espèces aux inégalités entre femmes et hommes. Les mesures que nous avons élaborés ensemble en bonne Intelligence s'inscrivent dans une lignée d'avancer que nous. Avons prises en faveur de la santé des femmes pour mieux garantir leurs droits reproductifs améliorer leur prise en charge spécifique renforcer le dépistage et la prévention. Je pense par exemple à la prise en charge à 100% pour toutes les femmes la contraception d'urgence à la gratuité des protections hygiéniques ou encore à la grande campagne de vaccination contre le papillomavirus des filles et des garçons qui débutera à la rentrée prochaine dans tous les collèges et qui nous permettra d'envisager la possible éradication du cancer du col de l'utérus. Le Parlement tient en la matière un rôle central. Je pense ici à certaines grandes lois. La loi Neuwirth de 67 autorisant la contraception, la loi Veil dépénalisant d'IVG en. 75 ou encore plus récemment la dernière loi de bioéthique autorisant la PMA pour toutes. Si ce qu'on veut qu'ici ces grands textes c'est parce que toute loi participant à combler les inégalités entre femmes et hommes toutefois participant à améliorer la santé des femmes toute loi permettant de redonner un peu plus la main sur leur corps et leur vécu et je le pense, une grande loi. Et le texte que nous allons adopter aujourd'hui, participe à sa manière, à ce grand combat. Je vous remercie. remercie Monsieur le Ministre, je rappelle qu'en application de l'article 42 alinéa à 12 du règlement, le Sénat statut par un seul vote sur l'ensemble du texte. Nous passons. Explications de vote, des groupes à raison d'un orateur par groupe. J'invite Monsieur Bernard Fiolet. Notre collègue du groupe RDSE à prendre la parole pour cinq minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, madame la présidente. Mes chers collègues. Quand la mort survient avant la naissance à n'importe quel stade de la grossesse, c'est très souvent une expérience éprouvante pour la femme mais également pour les partenaires. Si les fausses couches sont relativement fréquentes et bénignes. Beaucoup de parents se projette cependant très tôt dans une vie de famille. Et le secret qui entoure les 3 premiers mois de grossesse rend leur deuil encore plus difficile les abandonnant à la solitude de leur chagrin. D'autant qu'il existe toujours un tabou autour de la perte d'un bébé qui n'a jamais existé aux yeux des autres. Selon une étude de 2019, réunissant des chercheurs belges et britanniques près d'une femme sur six ça aurait ainsi victimes de stress post-traumatique, après une fausse couche au cours du 1er trimestre. Elles se sentent coupables ont le sentiment que leur capacité à être maire est remise en question et la plupart éprouve un sentiment d'échec et de vide. Pour autant. Les conséquences d'une interruption spontanée de grossesse sont encore trop souvent minimisé voire ignoré. Le professeur René Frydman parle même d'un vide juridique et souligne qu'il n'existe actuellement en France aucun protocole aucun parcours ni réseaux organisés. Pour répondre à la demande des coups d'explication d'orientation de ces couples en détresse. C'est ce à quoi on tend répondent cette proposition de loi. Elle permet de reconnaître la douleur et les besoins spécifiques de ces couples et met en place des mesures concrètes en vue de leur apporter le soutien nécessaire pour traverser cette épreuve et se reconstruire émotionnellement. Les travaux tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat ont permis d'enrichir ce texte. Il est ainsi prévu que chaque ARS mettent en place un parcours spécifique médical et psychologique pour mieux informer et orienter les patientes comme leurs partenaires de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont vécu une fausse couche. Le Sénat a introduit une protection contre le lit 600 le licenciement pendant les 10 semaines qui suivent une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu entre la 14ème et la 21ème semaine d'aménorrhée. Surtout. Nous nous félicitons de la suppression du délai de carence désormais les femmes qui font d'une fausse couche pourront bénéficier d'un arrêt de maladie indemnisés dès le 1er jour. Et cette mesure concernera les salariés mais aussi les fonctionnaires les indépendante et les non-salariés agricoles. Cette proposition de loi permettra également aux sages-femmes d'adresser leurs patientes et leurs partenaires à un psychologue conventionné, dans le cadre du dispositif mon parcours psy. Cette prise en charge psychologique me semble essentielle car elle permet de reconnaître la détresse de ces couples et de leur offrir le soutien dont ils ont besoin. Pour autant. Nous pouvons nous interroger sur l'efficience de ce dispositif créé en avril 2022, qui prévoit le remboursement par l'assurance maladie du 8 séances par an. Ah d'accompagnement psychologique de 30 minutes chez un psychologue conventionnés. Au bout d'un an. Mon parcours psy a en effet montré ses limites. 93%. Des psychologues ont refusé de s'y inscrire de s'inscrire sur la plateforme et seulement 90.000 vous avez dit, 130.000 patients ont bénéficié du dispositif. Dans ces conditions on peut craindre que les coupes confrontés à un tel drame ne puisse finalement pas d'y accéder. C'est pourquoi nous nous félicitons que la CMP et conserver l'article 1er bis a introduit au Sénat sur proposition d'Annick Billon et de notre collègue, Véronique Guillotin. Il s'agit d'étendre le Champ d'un rapport sur l'accessibilité de mon parcours psy prévue dès la mise en place du dispositif. Afin qu'il étudie spécifiquement l'accès des couples confrontés à une fausse couche aux séances de suivi psychologique, prise en charge. Nous ne pouvons pas prendre le risque de passer à côté des objectifs poursuivis par cette proposition de loi. Cette proposition de loi, Monsieur le Ministre. Monsieur le rapporteur, que nous allons voter. Avec. Sérénité. Si cher collègue, la parole est à présent à notre collègue la sénatrice Madame Florence là Sarah du groupe les républicains. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous allons nous prononcer sur les conclusions de la CMP sur la proposition de loi visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse dite fausse couche. Encore aujourd'hui, il existe une forme de tabous autour de la fausse couche. Les couples ne bénéficient d'aucun dispositif d'accompagnement, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'un non événement. Or une fausse couche, peut être un événement traumatisant. Qui affecte chaque femme différemment et peut entraîner de l'anxiété une dépression et même des symptômes, ça s'apparentant au stress post-traumatique. L'interruption spontanée de grossesse concerne près de 15% des grossesses. Selon une étude menée par le Collège national des gynécologues et hop stressé et obstétriciens français 200.000 grossesses s'arrêtent chaque année au cours des 5 premiers mois. Il était donc nécessaire d'essayer d'apporter des réponses à la prise en compte de la douleur des parents qui subissent une fausse couche. Le texte initial de la proposition de loi était centré sur le suivi psychologique des femmes, faisant une fausse couche. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui propose une prise en charge des couples qui englobe les questions de suivi psychologique, mais aussi d'information d'orientation et de suivi médical. Le Sénat, et plus particulièrement la commission des affaires sociales a pris toute sa part dans l'enrichissement de ce texte. Je tiens à cet égard, a salué le travail de notre collègue rapporteur Martin lévrier. Ainsi, ce texte prévoit la mise en oeuvre par les agences régionales de santé d'un parcours spécifique associant, médecins, sages-femmes et psychologue pour la prise en charge des interruptions spontanées de grossesse d'ici au 1er septembre 2024. L'information et le suivi médical et psychologique des des couples. Devraient être ainsi améliorer par ailleurs le texte otages davantage les femmes lorsqu'elles sont en activité en effet en cas d'arrêt maladie, le délai de carence et supprimé. On l'a dit, pour toutes les salariés indépendante et les travailleuses. Non c'est la non-salariés agricoles. Cette mesure permettra aux femmes de percevoir une indemnisation dès le 1er jour d'arrêt. Le texte prévoit également une protection de 10 semaines contre le licenciement au bénéfice de femme confrontée à une interruption spontanée de grossesse dite tardive médicalement constatée et Lyon lieu entre la 14e et la 22e semaine d'aménorrhée. Le groupe Les Républicains considèrent que ce texte contient des avancées qu'il convient de soutenir. C'est pourquoi nous voterons en faveur de ce texte. Merci cher collègue là. Parole est à présent à monsieur Claude Malhuret, monsieur le président du groupe des indépendants et vous avez 5 minutes, chers collègues.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

c'est encore davantage le cas lorsque le texte dont elle est l'objet vise à mieux accompagner les couples qui traverse une expérience difficile tels que la fausse couche. Événement qui touche environ 200.000 femmes par an dans notre pays et qui concerne une grossesse sur 4 les fausses couches sont malheureusement un phénomène fréquent. Cela était bien indiqué lors de nos échanges en commission. Mais je pense important de le rappeler une fois de plus. Il y a autant de façons de vivre une fausse couche, qu'il y a 2 femmes et bien sûr une même femme peut vivre bien différemment sa 2ème fausse couche de la 1er certaines peut ne pas le vivre comme un traumatisme, ni même comme une souffrance. D'autres peut le vivre comme un drame comme la perte d'un bébé qu'elles aimaient déjà. C'est évidemment surtout à ces dernières que ce texte s'adresse sans pour autant exclure les premières. Ce texte vise à proposer aux femmes et éventuellement leurs partenaires un accompagnement psychologique aujourd'hui assez rarement proposé. Un événement dit fréquent ne veut pas automatiquement. Dire qu'il est banal et encore moins pour celles qui le vit. La création d'un parcours dédié dans chaque ARS prévoit de coordonner tous les acteurs susceptibles d'intervenir dans la prise en charge des femmes victimes ne fausse couche tout comme développer la formation des médecins, des sages-femmes et des psychologues sur ce phénomène et systématiser l'information auprès Nous saluons. Grâce à un amendement du gouvernement, la suppression du délai de carence dans le cadre d'un arrêt maladie, faisant suite à une interruption spontanée de grossesse que nous trouvons être un point d'équilibre satisfaisant entre la création d'un congé spécial et la situation actuelle. Plus largement, l'adoption de cette disposition témoigne d'une meilleure prise en compte de la femme dans le monde du travail et des adaptations qui mériteraient d'être envisagée ou au moins discuter. Ces différents sujets. Montre que l'égalité entre les hommes et les femmes au travail ne se limite pas à la seule mais non moins importante question de l'égalité salariale, ouvre également la possibilité pour les sages-femmes d'adresser leurs patientes et leurs partenaires à un psychologue via le dispositif mon parcours, si c'est une mesure en totale adéquation avec le rôle et les compétences et Schramm actrice essentielle dans l'accompagnement des femmes enceintes. Si nous nous réjouissons de cette CMP conclusive c'est aussi car elle a maintenu quasi intégralement les améliorations que notre chambre avait apporté au texte l'extension tout à fait justifiée aux salariés ou non salariés agricoles et aux indépendante de la suppression du délai de carence sur les arrêts, faisant suite à une fausse couche et l'intérêt et l'instauration d'une protection. Contre le licenciement pendant 10 semaines après une fausse couche cela a été dit dans cette chambre comme à l'Assemblée nationale. L'efficacité de ce texte repose sur le dispositif mon parcours aussi dont on connaît l'accueil réservé qu'il a reçu de la part des professionnels. Si adoptée au Parlement un dispositif en faveur de l'accompagnement psychologique des femmes est un 1er pas. La véritable avancée sera de le rendre applicable et effectifs. Dans cette perspective, notre groupe votera en faveur de ce. Je vous remercie, cher collègue, la parole est à présent à madame Mélanie Vogel, du groupe des écologistes et vous avez 5 minutes, chers collègues. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Je tiens d'abord à remercier l'autrice de cette proposition. La députée Sandrine Josso, ainsi que notre rapporteur Martin lévrier pour tout le travail effectué l'examen a permis de discuter d'un sujet largement tabou dans notre société, celui des fausses couches, qui comme toutes les affaires dites de femmes ou plutôt comme toutes les affaires de corps des femmes ou plutôt je pense comme toutes les affaires de corps des femmes non sexuelle Isablle qu'on ne veut pas voir demeurent des sujets que l'on traite peu comme les règles qui concernent 15 5 millions de femmes et qui demeure aujourd'hui un sujet tabou, les fausses couches, qui concerne environ un quart des grossesses chaque année, soit 200.000 grossesses par an sont hein ce phénomène à la fois tout à fait normal et tout à fait mal géré. Ce tabou il est comme tous les tabous. Source de nombreux dysfonctionnements. On gère très mal ce dont on parle trop peu. C'est donc le rôle du législateur que de s'emparer de cette question et de s'en emparer avec en ligne de mire cette réalité, il y a au fond comme les règles comme les avortements comme tout ce qui touche à la santé reproductive, autant de cas que de personnes une fausse couche peut survenir dans le cadre d'une grossesse désirée mais aussi dans le cas d'une grossesse hein. Une fausse couche peut passer inaperçu. Une fausse couche peut être facilement vécu une fausse couche peut être physiquement éprouvante psychologiquement difficile et les deux à la fois une fausse couche là peut être terrible et ça peut aussi être pas pas chose et notre cadre juridique doit garantir que les personnes soient prises en charge et respecté dans tous les cas qu'elle souffre qu'elle ne souffre pas qu'elle soit soulagée qu'elle soit effondré à la manière dont elles le souhaitent. Notre cadre juridique doit aussi reconnaître que ce n'est pas qu'une affaire de femmes enceintes ou qu'en tout cas ça ne l'est pas toujours dans le cadre d'un projet parental à deux les deux personnes peuvent être touchées et touché différemment. Et c'est par la prise en charge juridique de cette réalité que l'on fera aussi progresser l'égalité des droits. Alors, avons-nous dans ce texte répondu aux anges. Le changement de terme déjà et à mon avis positif et à ne pas sous-estimer interruptions spontanées de grossesse c'est beaucoup plus juste que fausse couche, comme si quelqu'un avait commis une faute. La suppression du délai de carence pour les arrêts maladie consécutif à une fausse couche à une interruption spontanée de grossesse pardonnez-moi constitue une avancée concrète et importante. Tout comme l'amélioration de la formation des professionnels de santé qui est un impératif absolu au vu des récits qui sont toujours aujourd'hui, a rapporté. La protection contre le licenciement pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse est également une bonne chose. Toutefois, je déplore que ce texte reste largement en deçà des enjeux. introduit de congé spécial pour le couple confronté à une interruption spontanée de grossesse un tel congé. Et je veux le répéter ici fondée sur le choix sur la liberté de le prendre ou de ne pas le prendre aurait permis aux personnes concernées de se reposer de prendre un peu de temps pour elle et pour eux si elle le souhaite, d'autres pays ont mis en place avec succès un tel congé spécial, tout comme certaines entreprises en France aussi certaines personnes en France pourront donc en bénéficier et d'autres non, constituant ainsi une rupture manifeste je crois de l'égalité des droits. Je regrette. Également que le Sénat et supprimée l'1er bis de ce texte qui visait à créer un parcours de soins spécifiques. Par ailleurs, de manière générale, les effets de ce texte resteront limités dans le contexte d'un système de soins délaissé ou la grossesse est prise en charge de manière partiellement partiellement insatisfaisante. Un exemple, la prise en charge des frais liés à la grossesse comme l'avait proposé ma collègue Raymonde Poncet Monge. Il faudrait que l'ensemble des frais liés à la grossesse dès les premières semaines puissent être prises en charge par la Sécurité sociale.

Le dispositif mon parcours si. Pour rappel, ça a été dit plusieurs fois, ce dispositif était au coeur de ce texte, dont la seule et unique mesure était initialement de permettre aux maïeuticienne et maïeuticien d'adresser les patientes et patients psychologue pour des séances dans le cadre de mon parcours Or on le sait, ce dispositif s'avère défaillant comme les psychologues le juge inadapté aux besoins seulement 7% y participent. Vous l'aurez compris, nous considérons évidemment que ce texte comporte des avancées. Mais qu'il est bien loin de faire ce que son titre suggère accompagné véritablement les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse nous le voterons bien sûr mais nous rappelons. Nous appelons le gouvernement comme sur tant d'autres sujets a cessé de s'appuyer sur des PPL ici et là qui apporte régulièrement de petites touches améliore hâtive à notre système la santé sexuelle et reproductive est un grand sujet elles méritent une grande loi pour une prise en charge globale. Je vous remercie. Merci. La parole est à présent à Madame, Patricia Schillinger, du groupe RDPI vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En est saisissant de la situation des femmes victimes d'interruptions spontanées de grossesse dite fausse couche. Nous nous attaquons à un des nombreux tabous dont souffrent encore. Le corps de femme. au travers de monde propres combat contre la précarité menstruelle. J'ai pu observer comment notre société pouvait encore ignorer certaines souffrances Pesci figues aux gens féminin. Or cette ignorance discriminent et exclut. Aussi avec le groupe RDPI je me réjouis de l'accord sur lequel sont parvenus, députés et sénateurs lors de l'examen de cette proposition de loi en commission mixte paritaire. J'en profite pour saluer au passage le travail de Sandrine Josso, auteur de ce texte et rapporteur pour l'Assemblée nationale et la. Encore une fois, de s'être saisi de ce sujet important, le texte qu'initialement compter 2 articles a pu être enrichi au cours de la navette législative. Je salue à ce titre, le travail de notre rapporteure Martin lévrier qui, dans l'intérêt des premières concernées a su mener un dialogue constructif pour aboutir en bonne Intelligence. Ah un texte à la hauteur de ce, de cet enjeu de société. Je rappelle que ce sont en effet près de 200.000 fausses couches qui sont détectés chaque année en France, alors qu'entre 20 et 55% des femmes qui en sont victimes présentent des symptômes dépressifs et que 15% d'entre elles connaissent un état de stress post-traumatique, aucun accompagnement, aucune prise en charge ne leur est actuellement proposé ainsi la principale mesure de ces tests con texte consiste à proposer un un accouchement psychologique adaptés aux femmes dont la santé mentale peut être affectés par une interruption spontanée de grossesse. Le texte habilite. Pour ce faire, les sages-femmes à adresser leurs patients à un psychologue dans le cadre du dispositif mon parcours psy je ne plusieurs avancées importantes apportées par la navette parlementaire. L'extension de cet accompagnement au ou à la partenaire de la de la patiente et la reconnaissance du rôle du premier de 1er plan des sages-femmes dans la cour, l'accompagnement de la grossesse. Je salue également la suppression voulue par le gouvernement du délai de carence pour l'indemnisation des hein. Des arrêts de travail consécutifs à une interruption spontanée de grossesse de plus son extension aux travailleuses indépendantes et les non-salariés agricoles initiée par le rapporteur et bénéfique pour les, ces femmes, il s'agit en effet de permettre à toute de bénéficier de ce progrès en a les gens, notamment les contraintes financières que peut engendrer un arrêt de travail. Je tiens enfin à souligner l'engagement du gouvernement qui a tenu à protéger les femmes des discriminations professionnelles qui peut susciter le désir de parentalité révélé à la suite de la perte d'un foetus ainsi que les conséquences psychologiques que cela engendre la protection des femmes concernées s'inscrit dont légitimement dans ce texte. Notre groupe RDPI votera donc pour. Cette proposition de loi qui reconnaît, d'une part la souffrance des femmes victimes de fausses couches et d'autre part, propose un accompagnement nécessaire et soutenue aux couples concernés je tiens enfin à saluer une fois encore le travail réalisé par nos deux chambres et l'esprit transpartisan qui a caractérisé le travail législatif tout au long de cet examen texte. Cher collègue, la parole est à présent à Madame Émilienne. Pumerole du groupe socialiste et vous avez 5 minutes, chers collègues. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Chers collègues, je me félicite. Que le Sénat soit aujourd'hui réunis pour voter les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à améliorer l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse qu'on appelé donc autrefois fausse couche. En effet en sciences ici même au Sénat, nous avions tous souhaiter une mise en oeuvre rapide des dispositions de ce texte qui permettront une meilleure reconnaissance et une visibilité des interruptions spontanées de grossesse. Je le dit en préambule, ce texte un pas supplémentaire pour la santé des femmes ce qui justifie notre vote favorable et notre soutien aujourd'hui. En effet, grâce aux travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, le texte initial a été enrichi et le dispositif d'accompagnement étoffé. Je redis l'article 1er. Ah prévoit l'institution par les agences régionales de santé d'un parcours spécifique qui associera donc les médecins, les sages-femmes, les psychologues dans une prise en charge des interruptions spontanées de grossesse, il permettra d'améliorer l'information, le suivi médical, le suivi psychologique des patients et de leurs partenaires. Il permettra aussi de renforcer la formation des professionnels de santé, c'est important. L'article 1 B du texte supprime le délai de carence applicable aux arrêts maladie consécutif à une interruption spontanée de grossesse. Pour les assurés du régime général et assimilés, mais aussi pour les agents publics et pour les assurés des régimes spéciaux et je salue le travail du Sénat qui a élargi la suppression de ce délai de carence, quel que soit le statut des femmes aux travailleurs donc indépendant et non salariés agricoles aussi. L'article 6 qui a été ajoutée par amendement donc au niveau du Sénat instaure une protection de 10 semaines contre le licenciement pour les femmes qui sont confrontés à ce problème-là. Après la 14ème semaine d'aménorrhée. Cette mesure a pour but de lutter contre les risques de discriminations professionnelles dont les femmes sont malheureusement bien souvent victimes. Enfin, l'article 1er bis est également l'issue de nos travaux au Sénat Entend étendre chante d'un rapport sur l'accessibilité du fameux parcours psy afin qu'il analyse précisément l'accès des couples. Qui sont donc confrontés à ce problème aux séances de suivi psychologique qui sont pris en charge. Néanmoins, nous le saurions parler pour ce texte d'une réelle avancée très importante année fait nous ne pouvons que regretter que les sages-femmes ne puissent bénéficier de la capacité prescriptives et effectué un accompagnant médical des femmes victimes d'une interruption spontanée de grossesse. Alors que cette compétence leur que cette compétence leur est reconnu en cas d'interruption volontaire de grossesse et il s'agit là d'un parfait illogisme. Que je ne peux m'expliquer les sages-femmes étant une profession médicale, spécialisé dans la santé reproductive des femmes. De plus ne recruterait ton que notre proposition visant à mettre en place un congé spécial de 3 jours pour les femmes confrontées à l'interruption spontanée de grossesse n'ait pas été adopté ce congé crée un droit nouveau un droit du travail pour les femmes en leur laissant le choix et en particulier, notamment celui de ne pas. Dépendre de leur médecin pour bénéficier d'un temps de récupération nécessaires, je crois qu'elle pouvait prendre, donc oui ou non enfin. La proposition de loi ne renforce pas le dispositif. Mon parcours psy qui reste largement insuffisant. Monsieur le Ministre, vous le savez pour garantir le suivi psychologique des 200.000 femmes cela été évoque à plusieurs reprises qu'ils doivent faire face à une interruption spontanée de grossesse chaque année. Mises en place depuis plus d'un an des collègues dit 93% des psychologues ni à des repas. Seuls 7% ce bip dispositif n'a bénéficié n'ai pas les mêmes chiffre que vous Monsieur le Ministre, moi j'ai 76.375 76.375 mais en tout état de cause c'est peu même si c'est 130.000 comme vous l'avez évoqué, c'est peu et donc si cette proposition et nous l'avons dit. Une première étape vers la reconnaissance des interruptions spontanées de grossesse et plus généralement de la santé des femmes. Le chemin est encore long. Monsieur le ministre, il est désormais indispensable d'accompagner ces situations dans une approche holistique de la santé des femmes et de mettre enfin en place une politique publique globale de la santé sexuelle et reproductive des femmes. Merci. Merci cher collègue. La parole est à présent un notre collègue Madame Laurence Cohen du groupe communiste et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 1er juin dernier, la commission mixte paritaire a trouvé un accord sur cette proposition de loi visant, donc l'accompagnement des couples confrontés à une fausse couche. Nous saluons l'esprit transpartisan qui a guidé les modifications apportées au texte tout au long de ce de son cheminement parlementaire et qui permettent de contribuer, de lever le tabou des fausses couches vécu chaque année par 200.000 femmes dans notre pays et qui concerne près de 15% des grossesses et donc autant de concubins et de concubines, nous sommes partis d'un dispositif centré sur le suivi psychologique des femmes, faisant une fausse couche pour arriver à un parcours qui s'adresse aux couples et englobe les questions de suivi psychologique également d'information d'orientation et de suivi médical désormais le jour de carence sera supprimée pour tous les salariés indépendants et travailleurs non salariés agricoles. Le Sénat instaurer une protection de 10 semaines contre le licenciement au bénéfice des femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse tardive après la 14ème semaine d'aménorrhée, il aurait sans doute mieux valu l'étendre à un stade plus précoce de la grossesse, la douleur due à la perte d'un enfant n'étant pas fonction du nombre de semaine d'aménorrhée néanmoins ces disposition améliore sensiblement les garanties prévues par le code du travail visant à protéger les femmes contre les risques de discrimination professionnelle. Je rappelle qu'en matière de droit du travail depuis 2016 l'obligation de surveillance médicale renforcée de la femme enceinte a été remplacé par un suivi médical renforcé pour lequel l'état de grossesse n'est plus pris en compte en tant que telle l'obligation de suivi individuel renforcé pour toutes les femmes enceintes relève donc d'une nécessité en droit du travail. Enfin sur le coeur du dispositif qui concernent l'accompagnement psychologique des patientes et de leurs partenaires nous redisons ici comme en première lecture que nous avons de sérieux doutes. Monsieur le Ministre, sur la capacité du dispositif bon parcours psy à répondre aux enjeux et nous avons été plusieurs dans l'hémicycle à le faire. Vous voulez étendre aux couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse un dispositif auquel seulement 13% des psychologues ont fini par adhérer temps cet outil suscite la colère de la profession selon le rapport d'information sur le printemps social de l'évaluation, 2023. Coécrit par d'autres collègues député Pierre Dharréville mon parcours psy présente plusieurs défauts de conception. Tout d'abord le faible nombre de prise en charge. La tarification des séances qui ne sont pas suffisamment attractive. Ensuite, les conditions d'adressage préalable par ingénieur réaliste alors que 6 millions de nos concitoyennes et de nos concitoyens n'ont pas de médecin traitant et conditions qui induisent donc une mise sous tutelle médicale des psychologues. Enfin les critères d'éligibilité des patients qui sont inopérant et inadapté par ailleurs mon parcours psy a été présenté par le gouvernement comme un outil d'accès aux soins psychiques, avec un remboursement par l'assurance maladie à hauteur de seulement 60% et les 40% par les complémentaires santé. Monsieur le Ministre, les chiffres démontrent que le dispositif est non seulement rejeté par la majorité des psychologues, mais qu'en plus il a raté sa cible puisque seulement 10% des précaires sont entrés dans le dispositif. Comme j'avais eu l'occasion de vous le dire déjà en première lecture cette vision comptable de la prise en charge de la santé mentale s'oppose à la fois à la réalité de la prise en charge globale des patients, mais également à la situation économique des Françaises et des Français, dont près de 3 millions ne dispose pas de complémentaire santé ni d'ACS. Quand allez-vous donc entende les revendications des psychologues et abroger ce dispositif mon parcours si Monsieur le Ministre, ou tout de moins quand allez-vous ouvrir de véritables négociations avec cette profession qui rejettent ce dispositif. En conclusion, même si nous regrettons le rejet de notre amendement pour associer les sages-femmes à cet accompagnement des fausses couches et celui pour créer un congé de trois jours pour les couples concernés, comme cela existe depuis 2021 en Nouvelle-Zélande. Mon groupe, le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste votera en faveur de cette. Proposition de loi. Je vous en remercie donc. Unanimité sur le vote mais avec quand même hein on attire votre attention sur un certain nombre de choses. Merci. Si cher collègue. La parole est enfin à madame Brigitte de visas du groupe Union centriste et vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avant tout, je tenais à saluer monsieur le sénateur Martin lévrier pour la qualité de son rapport la teneur des échanges en commission mixte paritaire et l'accord qu'il a pu obtenir avec les sénateurs et les députés qui composé la CMP et j'en profite également pour saluer Madame la députée Madame je chaussant pour le texte que vous avez sur lequel vous avez travaillé. Merci. Alors s'il est à noter que le Parlement a su trouver un accord constructif transpartisan traduisant le caractère unanime autour de cette proposition de loi ou du moins témoignant d'un soutien global pour ce texte, les suggestions, les problématiques soulevées par l'Assemblée nationale et par le Sénat met en lumière l'attente de positionnement de la part du gouvernement appelé à travailler la question de l'accompagnement hospitalier de manière plus assidue plus concrètes. L'implication des sages-femmes dans le processus d'accompagnement des couples dont découle la question de leur formation, mais de leur statut, de leurs nombres de la rémunération et de leur reconnaissance n'est pas traité de manière suffisamment sérieuse. Des voix se sont aussi levé pour exprimer l'insuffisance du texte pour améliorer l'accès à l'information et au suivi psychologique. La situation matérielle, économique des structures du monde médical et hospitalier dans notre pays doit être réfléchi dans son intégralité les efforts récents ne compense pas les rationalisations du passé. Notre système de santé doit être soutenu et ce soutien passe par la confiance envers les professionnels de santé. Ceci étant dit, Monsieur le Ministre, nous pouvons nous réjouir collectivement des avancées apportées par cette loi. Je pense qu'à la suppression du délai de carence pour l'indemnisation des congés maladie liées une interruption spontanée de grossesse ou encore la protection contre le licenciement pour les femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse tardive. Le travail du Sénat a permis de renforcer les objectifs d'information a signé au parcours et renommé le parcours de fausse couche en interruptions spontanées de grossesse par une terre le terminologie plus médicalement précise et moins stigmatisante et de populariser le terme encore trop peu utilisé. Retenons aussi l'instauration d'une protection de 10 semaines contre le licenciement pour les femmes confrontées et interruptions spontanées de grossesse tardive visant ainsi à limiter les effets de seuil et à prévenir les discriminations. Professionnelles je regrette par ailleurs que le Sénat n'est pas retenu la proposition de l'Assemblée nationale, demandant un rapport sur l'extension de l'assurance-maternité dès les premières semaines d'aménorrhée, jugé trop complexe sur le plan opérationnel. Il était temps que dans notre pays un protocole existe, nous l'avons dit lors de nos travaux, environ 200.000 femmes sont concernées chaque année par une interruption spontanée de grossesse dans notre pays une grossesse sur 4 se termine en moyenne par une une interruption spontanée de grossesse. Évidemment, sur certaines femmes sûrement de cet aléa, d'autres le vivre de manière dramatique individuellement ou en couple, je me je réjouis que cette proposition n'est pas oublier les compagnes et compagnons des femmes affrontant ces situations. Je pense personnellement que cette proposition de loi visant à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse ouvrira la voie dans notre pays a une réflexion à un débat qui, qu'on le veuille ou non, se posera, quelle place pour le couple lors d'une interruption volontaire de grossesse. Derrière cette question, quelle place pour l'homme quelle reconnaissance quel accompagnement lors d'un IVG. La question est encore tabou mais en légiférant et en votant ce matin pour la combattre l'accompagnement du couple et non seulement l'accompagnement des femmes dans le processus de grossesse. Nous savons que nous ouvrons ou du moins que nous approfondissant un débat sociétal plus large. Cette proposition de loi n'est pas une fin à l'étau un commencement aussi notre groupe votera favorablement ce texte. Je vous remercie. Merci Charles. Collègues conformément à l'article 42 alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient. Cette proposition de loi est définitivement adoptée et à l'unanimité en ce qui concerne au Sénat. Merci cher collègue. informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur la proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des élus locaux dans la mise en oeuvre de la lutte contre l'artificialisation des sols ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. Mes chers collègues, je vais suspendre la séance elle sera reprise à 14h 50 pour la suite de l'examen du projet de loi de programmation mais il lit de terre. La séance est suspendue.